Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, maires se tient cette semaine, la proposition de loi que je vous présente aujourd'hui a pour but de faire passer un message clair et fort aux élus locaux, notamment à ceux de nos territoires ruraux le Sénat vous accompagne et soutient pleinement votre engagement précieux et vos initiatives en faveur du maintien des services de proximité. a prononcée la semaine dernière à destination de la presse régionale et des télévisions locales, le président Gérard Larcher a rappelé que le Sénat, « assemblée des territoires », se tenait aux côtés et au service des élus locaux. Cette proposition de loi s'inscrit ainsi pleinement dans une démarche volontariste d'aménagement du territoire. Elle part d'abord d'un double constat le sentiment d'abandon très fort de nos concitoyens en zone rurale, qui se conjugue à une certaine forme de solitude ressentie par les élus locaux face à un problème très concret de désertification bancaire. contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, il existe un réel problème de désertification bancaire en France. Qui, dans cet hémicycle, n'a pas sur son territoire l'exemple d'une agence ou d'un distributeur automatique de billets venant de fermer ou restant sous la menace d'une fermeture ? Un état des lieux de la Banque de France sera publié en 2019 qui établira une cartographie des zones de désertification bancaire. Toutefois, nous avons déjà une idée très précise de la tendance selon la Banque centrale européenne, 2 000 distributeurs automatiques et 300 agences ont disparu entre 2015 et 2016. Et les prévisions sont encore plus pessimistes d'ici à 2020, le groupe BPCE prévoit la fermeture de plus de 400 agences, quand la Société Générale a confirmé la réduction de 20 % de son réseau d'agences, soit la fermeture de 450 établissements en deux ans. De son côté, BNP Paribas a déjà fermé 236 guichets depuis 2012. Face à ce constat, de nombreuses initiatives locales ont vu le jour ces dernières années, entraînant la signature de conventions entre communes et établissements bancaires pour le maintien de distributeurs automatiques de billets, ou DAB. Ce sont précisément ces initiatives qui sont à l'origine de la présente proposition de loi, ainsi que les difficultés exprimées par les maires, confrontés à de nombreux refus des banques, à une prise en charge périlleuse pour leurs finances locales et à leur solitude extrême, liée à l'absence de soutien de l'État. Comme l'indique le titre de la proposition de loi, l'accent est mis sur les zones rurales, non qu'elles soient les seules concernées, mais pour la simple raison que leurs difficultés sont bien spécifiques et justifient des mesures d'urgence. Les territoires sont par nature inégaux, comme le soulignaient nos collègues sénateurs Louis-Jean de Nicolaÿ et Hervé Maurey dans leur excellent rapport de 2017. En milieu rural, le phénomène de désertification est grandissant et fragilise encore davantage certains territoires manque de médecins, de transports collectifs, couverture numérique et téléphonique défaillante, voire inexistante, absence ou fragilité des commerces de proximité Une partie de la population vit mal la disparition des services publics, mais aussi des services au public et des équipements utiles au quotidien. Ce ressenti, c'est aussi ce qui conduit à la colère et aux extrêmes. Je veux donc, à travers cette proposition de loi, rappeler qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone, qu'il n'y a pas de territoires de seconde zone. Exactement ! Nous, parlementaires, représentants de la République et des élus, devons être présents pour accompagner les territoires dans les grandes transitions et les grands défis de demain. Très bien ! Selon une étude de publiée en octobre 2018, l'attractivité des campagnes françaises est conditionnée notamment par la présence de services de proximité. derniers sur tous les territoires constitue une étape essentielle. Pour ce faire, plusieurs facteurs propres à la ruralité doivent être pris en considération. d'une part, à la présence de populations plus fragiles, vieillissantes et moins mobiles. Ces populations sont parfois dépendantes des espèces pour le règlement de leurs achats, et souvent dépendantes de leur voiture pour tous leurs déplacements. Faire plusieurs kilomètres pour retirer de l'argent constitue donc une difficulté supplémentaire, notamment pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, qui sont les premières victimes du désengagement des banques sur nos territoires. D'autre part, nos aînés s'approprient moins les moyens de paiement modernes et sont moins bien dotés en outils numériques. Il n'est pas question de nier l'émergence de nouvelles pratiques qui se portent davantage vers les outils et modes de paiement numériques. Mais considérer que la dématérialisation est aujourd'hui actée et bien vécue par l'ensemble de la population constitue, selon moi, une erreur fondamentale. Enfin, j'en viens à un argument majeur en faveur du maintien des distributeurs de billets : nos territoires ne bénéficient pas tous de la couverture numérique indispensable à l'utilisation d'un terminal de paiement électronique. Dans certaines zones où l'accès à internet et même à la téléphonie fixe est entravé, le règlement par carte bancaire se révèle tout simplement impossible. Que dire alors aux commerçants de centres-bourgs, qui n'ont d'autre solution que d'accepter les seuls règlements en espèces ? Puisque l'État, et le Sénat, s'engagent pour la revitalisation des centres-bourgs, lutter contre la désertification bancaire me semble une étape importante. Les distributeurs automatiques sont indispensables pour l'inclusion sociale de nombreux citoyens et vitaux pour les commerces de nos centres-villes. Deux propositions vous sont donc faites, mes chers collègues. La première s'adosse aux conventions passées entre les communes et les banques, en leur donnant un cadre juridique et en leur offrant un financement propre, reposant non plus uniquement sur les collectivités, mais sur un fonds alimenté par les contributions des banques et piloté par la Caisse des dépôts Des réserves ayant été émises quant à la participation financière de la Caisse, nous présenterons un amendement visant à l'en exclure. Concernant la gestion du fonds, la Caisse des dépôts s'y est montrée plutôt favorable, indiquant qu'il s'agissait précisément de son coeur de métier. La seconde proposition vise à renforcer le maillage territorial, l'introduction d'un critère de distance minimale des bureaux de poste dotés de DAB. Cette disposition semblant poser des difficultés techniques et financières, nous laisserons le débat parlementaire trancher. Madame la rapporteur, votre rapport décrit parfaitement la situation actuelle et les difficultés grandissantes sur certains territoires. Notre constat est le même. Toutefois, nous avons quelques divergences sur les solutions à apporter. À l'article 1, qui concentrera l'essentiel des débats, services, l'artisanat et du commerce, le FISAC, à l'aide à l'installation de distributeurs de billets dans les commerces, en zone blanche uniquement. C'est une bonne idée ! Cette proposition fait encore peser sur le budget de l'État, et sur les commerçants, les défaillances des banques, d'autant plus que la pérennité du FISAC est loin d'être assurée. De notre côté, nous considérons que le fonds de maintien et de création de DAB doit être alimenté par les banques, une fraction du produit de la taxe dite « emprunts toxiques », procédant d'une logique de responsabilisation sociale et territoriale des banques.

est subordonnée à une couverture numérique stable et à la bonne volonté des commerçants. Or, d'une part, ces derniers n'y sont pas nécessairement favorables, car ils seraient prélevés pour assurer un service bancaire et pallier le désengagement des établissements bancaires, et, d'autre part, ils ne sont pas ouverts en continu. Enfin, la souplesse du dispositif permettrait une adaptation de la réponse en fonction des territoires. Les demandes seraient étudiées au cas par cas par le conseil de gestion du fonds, qui déterminerait le montant total de la subvention dans le temps, sur la base des règles de calcul précisées par décret. Pour le reste, j'y reviendrai lors de la discussion des articles. Comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas question de nier ni de déplorer la dématérialisation croissante des moyens de paiement. Il est question de rappeler que celle-ci ne profite pas à tous, notamment en zone rurale, où la perte des services bancaires se fait particulièrement ressentir. Pour cette raison, et pour la réalisation concrète de l'égalité entre territoires, l'enjeu majeur de ces prochaines années demeure l'inclusion numérique. Nous avons adopté il y a peu la proposition de loi, déposée par le groupe du RDSE, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires et avons débattu de l'intégration, au sein de cette dernière, de l'Agence du numérique. Si nous souhaitons cette intégration au plus tôt, c'est précisément pour permettre une couverture numérique de tous les territoires dans les plus brefs délais. Dans cette attente, la présence de distributeurs de billets demeure indispensable. C'est pourquoi je soumets au débat parlementaire cette proposition de loi de transition, en espérant vivement que, demain, la couverture numérique de l'ensemble des territoires permettra à tous de bénéficier des mêmes outils de paiement et ne laissera personne, commerçant ou client, quels que soient leur lieu d'habitation et leur degré d'inclusion numérique, au bord du chemin. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, Éric Gold a rappelé le cadre et les objectifs de sa démarche. Je souscris à ses constats, car, quelles que soient les caractéristiques de nos territoires, nous sommes tous confrontés à une dévitalisation progressive. Pour autant, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de fatalité et qu'une action résolue et conjointe permettra d'enrayer ce phénomène. La proposition de loi contient deux solutions complémentaires à chacun de ses deux premiers articles, le troisième étant classiquement dévolu au gage sur les tabacs. L'article 1 prévoit la création d'un fonds dédié au maintien et à la création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales. L'article 2 étend la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste, en prévoyant que chacun de ses 17 000 points de contact doit comprendre un distributeur automatique de billets. Cependant, juridiquement, le mécanisme proposé n'est pas opérant. En effet, il est proposé la création d'un fonds c, financé essentiellement par l'affectation d'une part des ressources du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant conclu des emprunts à risque. Or les ressources de ce fonds ont été calibrées afin de répondre aux demandes qui lui ont été soumises. Nous le savons tous, le fonds de soutien joue un rôle essentiel pour les collectivités concernées il ne saurait être question de le réduire. La taxe qui l'abonde devrait être augmentée, ce qui n'est pas prévu par la proposition de loi. Par ailleurs, l'abondement envisagé du fonds n'est juridiquement pas possible. Il s'agirait de prélever une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ZE du code général des impôts- en clair, de réaffecter une part de la taxe dévolue à la résorption des emprunts toxiques souscrits par les collectivités. aux lois de finances du 1 août 2001 précise que « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances. Il est donc impossible, dans le cadre de la présente proposition de loi, de réaffecter une taxe déjà fléchée. Les ressources du fonds dont la création nous est proposée ne sont donc pas assurées. Éric Gold a rappelé qu'il nous revenait de répondre aux difficultés constatées dans les territoires et que notre débat résonnait particulièrement en cette semaine de Congrès des maires. Je partage son point de vue et j'ajoute qu'il nous appartient également de répondre concrètement Je souhaite rappeler quelques éléments chiffrés concernant l'activité bancaire. Notre pays compte plus de 56 000 distributeurs, répartis sur 14 000 communes. Depuis 2011, la baisse du nombre de retraits en espèces s'élève à 6 % : elle est supérieure à la diminution du nombre de DAB, qui est de 4,1 %. Parallèlement, les paiements par carte bancaire ont augmenté de 43 % ; ils représentent un volume de 10,5 milliards d'euros en 2017. Cette hausse résulte à la fois de coûts en baisse, permettant de payer par carte dès 1 euro, et d'une commodité accrue par le « sans contact », pour lequel le volume de paiements a été multiplié par cinq entre 2015 et 2017. Les paiements sans contact représentent désormais 10 % du volume de paiements par carte bancaire. Actuellement, les 6 305 agences postales communales peuvent délivrer jusqu'à 350 euros en espèces par semaine les 2 746 relais postes commerçants, jusqu'à 150 euros en espèces par semaine. Certains établissements bancaires ont déjà signé plus de 4 000 conventions avec des commerçants pour qu'ils installent dans leurs locaux des distributeurs automatiques de billets. Nous attendons la sortie du décret relatif au « », qui permettra aux commerçants de délivrer des espèces à l'occasion d'une opération pour l'achat d'un bien ou d'un service. L'implantation d'un distributeur automatique de billets coûte environ 90 000 euros et son entretien annuel, de l'ordre de 14 000 euros. Pour autant, ces révolutions des usages posent des difficultés à certains de nos compatriotes, pour des raisons territoriales ou générationnelles. Une réponse immédiate est donc nécessaire pour assurer l'égal accès aux espèces pour tous.

Lors des auditions que j'ai conduites, il m'a été indiqué qu'un groupe de travail sur l'accessibilité aux espèces avait récemment été mandaté par la Banque de France. Ce groupe de travail doit recenser l'offre d'accès aux espèces, tous canaux confondus, et définir les scénarios d'organisation de la distribution permettant de garantir l'accessibilité des espèces. Ce travail est complexe, compte tenu de la multiplicité des modes d'accès aux espèces. Aux côtés des distributeurs automatiques de billets des établissements bancaires existent également des distributeurs dans des commerces- il s'agit des 4 000 points relais -, les services postaux sans doute dès la fin de cette année, le « ». C'est à partir de ces différents outils que le groupe de travail doit remettre une cartographie en janvier prochain. Ce diagnostic mettra en évidence les situations de défaillance. Il sera alors indispensable qu'acteurs publics et privés locaux définissent une solution, à partir de la palette d'outils que j'ai mentionnée. J'ai rencontré MM. Philippe Wahl et Rémy Weber, présidents respectifs de La Poste et de La Banque postale, qui m'ont assurée de leur volonté de combler les éventuels manques sur le territoire. Je mets en garde, par ailleurs, sur l'effet pervers qu'engendrerait la constitution d'un fonds pour maintenir les DAB : il ne faudrait pas que les banques se mettent à exiger le recours à ce fonds pour rester sur nos territoires C'est pourquoi j'ai proposé, au nom d'une position pragmatique et réaliste, de pallier les situations de carence par un recours au FISAC. Ce recours serait réservé aux communes situées en zone blanche, car, pour les autres, le doit apporter une réponse supplémentaire.

cet amendement est indispensable : je vous invite à le voter en séance publique, le 30 novembre prochain. Surtout, je considère que cet amendement répond aux deux exigences qui doivent guider nos travaux identifier et relayer les problèmes constatés, et y apporter une réponse solide juridiquement. J'en viens à l'article 2 de la proposition de loi et à l'extension de la mission d'aménagement du territoire de La Poste. Cette évolution ne me paraît pas souhaitable, car je ne suis pas certaine que tous les maires se réjouissent à l'idée d'installer un DAB dans leur agence postale communale. De surcroît, le jeu de la libre concurrence pourrait paradoxalement conduire La Poste à héberger des distributeurs automatiques de billets d'un établissement bancaire concurrent de La Banque postale

Madame la présidente, monsieur le sénateur Éric Gold, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la lutte contre les déséquilibres au sein de nos territoires est une préoccupation centrale du Gouvernement. Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement a voulu conduire une action globale, transversale et mieux coordonnée en matière de cohésion territoriale et de cohésion sociale. Je n'en citerai que quelques exemples, qui sont bien connus des membres de cette assemblée : le programme « Action coeur de ville », par lequel 222 villes moyennes vont conclure un contrat de partenariat avec l'État et ses partenaires privés et publics pour la rénovation de leurs coeurs de ville le déploiement du numérique dans les territoires, grâce au plan France Très haut débit, pour permettre un accès au haut débit de qualité dans tous les territoires d'ici à 2020 et leur couverture en très haut débit d'ici à 2022

Je pense à la couverture en téléphonie mobile de qualité, qui sera généralisée dans les cinq prochaines années grâce à l'accord historique signé par les opérateurs de téléphonie mobile en janvier dernier. Mais c'est aussi, et l'auteur de la proposition de loi a raison de le souligner, l'accès aux services bancaires, notamment l'accès aux espèces et aux moyens de paiement.

Permettre l'accès de tous aux espèces, y compris dans les territoires ruraux, est donc un objectif tout à fait légitime. Au reste, il me semble compatible avec le souhait du Gouvernement de créer le meilleur écosystème possible pour développer des solutions de paiement innovantes. permettez-moi de rappeler quelques éléments factuels sur la couverture de notre territoire en services bancaires, notamment en matière de fourniture d'espèces. Alors que les espèces connaissent un recul progressif sur le plan du nombre de transactions réalisées, la France dispose toujours d'un maillage de distributeurs dense et de bonne qualité, environ 56 650 machines sur notre territoire. Selon la Banque de France, 87 % des habitants vivent à moins de cinq kilomètres d'un distributeur automatique de billets, et 98 % à moins de dix

Il est vrai, comme Éric Gold l'a souligné, que certaines banques ont entrepris de réduire le nombre de distributeurs. Mais il s'agit le plus souvent d'une rationalisation en zone urbaine, et ce n'est pas le choix de toutes les banques. Surtout, de nombreuses initiatives existent déjà pour favoriser un meilleur accès des territoires ruraux aux espèces, en complément des distributeurs automatiques de billets ou des guichets de banque sur nos territoires. Je pense, par exemple, aux points relais, qui permettent aux clients d'une banque de retirer des espèces auprès d'un commerçant, lequel agit comme agent bancaire par le biais d'une convention. Le développement de services bancaires proposés par les buralistes est également un exemple de l'inventivité des acteurs privés pour répondre aux besoins des citoyens. En l'occurrence, ces derniers peuvent ouvrir un compte bancaire auprès des buralistes qui le proposent. Du côté public, La Banque postale est un acteur majeur au service des populations rurales les plus isolées. Je rappelle que La Poste est chargée par la loi d'une mission de service public de contribution à l'aménagement du territoire, qui impose la présence d'au moins 17 000 points de contact sur l'ensemble du territoire. À ce titre, La Poste maintient, au-delà de ses besoins commerciaux, un réseau de points de contact dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d'outre-mer. Ces points de contact offrent un accès aux services financiers et au retrait d'espèces. La Banque postale dispose à ce jour d'un maillage robuste de distributeurs automatiques de billets : ces derniers sont près de 8 000, implantés dans près de 3 000 communes ou arrondissements de communes, dont 1 260 dans les communes rurales, en zone de montagne ou de ou de revitalisation rurale. Un Fonds postal national de péréquation territoriale, alimenté chaque année, pour la période 2017-2019, à hauteur de 174 millions d'euros par des abattements de fiscalité locale, permet notamment de financer le maintien de ce réseau. Ainsi, si je partage pleinement le souhait de garantir une accessibilité aux services bancaires de base pour tous nos concitoyens, y compris et surtout dans les territoires ruraux, je recommanderai volontiers

problèmes. Pour les banques qui possèdent déjà des distributeurs en zone rurale, ce dispositif de subvention créera un important d'effet d'aubaine. Il paraît très difficile de discriminer cette aide pour l'attribuer aux distributeurs non rentables,

Dans les zones qui ne disposent pas d'un accès aisé aux espèces, il n'est pas sûr que l'installation d'un DAB offre la solution la plus pertinente. C'est notamment le cas lorsqu'aucune banque n'est solidement implantée dans ce territoire, qui ne trouvera aucun intérêt à investir dans des équipements déconnectés de sa stratégie commerciale.

Au-delà de ces difficultés pratiques, ce dispositif pose en outre une importante difficulté juridique, notamment au regard du droit européen en matière d'aides d'État. Les ressources de ce fonds, en partie publiques, pourraient constituer une aide aux banques non conforme aux traités européens. De même, le fait que la loi confie, de manière unilatérale, la gestion d'un fonds à la Caisse des dépôts et consignations pourrait se révéler fragile du point de vue du droit de la commande publique. La gestion d'un fonds peut en effet s'analyser comme une prestation de services, qui doit donner lieu à une passation de contrat selon les règles du code des marchés publics. Enfin, j'émets des réserves sur la viabilité du dispositif au regard du droit budgétaire. Je souhaite ainsi rappeler qu'il n'est pas possible de mobiliser l'affectation d'une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ZE du code général des impôts. le produit de cette taxe est en effet affecté au fonds de soutien destiné à désensibiliser les emprunts à risque des collectivités locales. Par ailleurs, une telle mesure, qui serait de nature à créer de nouvelles charges non compensées pour l'État, ne pourrait figurer que dans une loi de finances. finances. En outre, la contribution éventuelle de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait résulter que d'une décision de cette institution, sauf à ce que le législateur choisisse de créer une charge non compensée pour la Caisse des dépôts Enfin, le dispositif de l'article 2, qui prévoit d'étendre la portée des obligations que la loi impose déjà à La Poste dans le cadre de sa mission d'accessibilité, aurait des effets déstabilisateurs pour les équilibres économiques de ce groupe, alors

il me semble prioritaire d'affiner notre diagnostic pour mieux cibler notre action. Comme vous l'avez noté, la Banque de France a engagé une cartographie de la desserte en espèces sur le territoire national. Ce travail de diagnostic nous permettra d'identifier précisément les zones où notre attention doit se porter prioritairement. Plus largement, nous suivons de près les évolutions de la filière des paiements pour continuer à garantir la disponibilité des espèces partout sur le territoire. Deuxièmement, il est indispensable de diversifier notre palette d'outils pour permettre une couverture aussi large et efficiente que possible du territoire en solutions de paiement.

Ce nouveau service offre également aux commerçants un moyen de gérer plus efficacement les encours en caisse. Les associations de commerçants ont unanimement souligné leur intérêt pour un tel service. Le décret d'application sera pris avant la fin de l'année, et je ne peux qu'encourager les citoyens et les commerçants à s'en saisir.

Le Gouvernement finalise actuellement la publication des textes d'application qui permettront le déploiement très rapide de cette solution d'accès aux espèces. Je note que certaines enseignes de la grande distribution ont d'ores et déjà lancé leur offre sur le fondement des dispositions législatives que vous avez votées. Il existe importante que nous devons poursuivre : le développement de solutions de paiement dématérialisées. Je rappelle que nous avons fortement progressé dans l'équipement des commerces en terminaux de carte bancaire. En France, plus de la moitié des transactions scripturales sont d'ores et déjà réalisées par carte, proportion supérieure à celle des paiements par carte dans la moyenne de l'Union européenne. Ce mouvement est appelé à se poursuivre. Le paiement sans contact connaît un véritable essor et offre une solution aisée pour le paiement de dépenses de la vie quotidienne d'un montant limité. Nous avons l'ambition d'aller plus loin dans le développement de ces technologies qui facilitent la vie de nos concitoyens et ne sont nullement réservées aux seuls citadins. Le développement du paiement en ligne ou du paiement par le biais de virements instantanés est également prometteur. Grâce au plan très haut débit et aux engagements du Gouvernement en faveur d'une couverture de téléphonie mobile de qualité, nous nous donnons les moyens de rendre ces technologies innovantes accessibles Enfin, le Gouvernement souhaite rappeler son attachement à la pérennisation de la mission d'accessibilité bancaire de la Banque postale sur tout le territoire. J'ai échangé ce matin même avec Philippe Wahl, président-directeur général de La Poste, qui m'a affirmé son engagement constant en faveur de cette mission. Les engagements réciproques Les engagements réciproques de l'État et de La Poste pour les quatre missions de service public qui sont confiées à cette dernière- service universel postal, contribution à l'aménagement du territoire, transports et distribution de la presse, accessibilité bancaire -font l'objet d'un contrat d'entreprise. Je réunirai vendredi prochain le comité de suivi de haut niveau de ce contrat d'entreprise avec l'ensemble des parties prenantes, dont le PDG de La Poste et les sénateurs Yvon Collin et Patrick Chaize. Nous aborderons à cette occasion du rôle de La Poste et de la Banque postale en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion bancaires, puisqu'il s'agit de la thématique qui a été retenue pour cette réunion. Nous demeurerons très vigilants sur ce

Au-delà de la création d'un grand pôle financier public, le rapprochement de La Poste avec la Caisse des dépôts et consignations permettra à ces deux groupes de combiner leurs forces pour assurer leur mission de service public en matière d'aménagement du territoire, ainsi que leurs interventions pour le développement économique territorial. Aussi, vous l'avez compris, je ne serai pas en mesure de donner un avis favorable à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Je propose en revanche de substituer au dispositif prévu à l'article 1 la conduite d'un diagnostic approfondi, qui prendrait la forme d'un rapport du Gouvernement ... Un rapport ! ... portant sur la couverture effective du territoire en solutions de paiement et d'accès aux espèces, et qui ferait le point sur la mise en oeuvre des différentes réponses que j'ai évoquées. Tel est le sens de l'amendement que je déposerai à l'article 1. Nous apporterons par ailleurs notre soutien aux amendements de suppression des articles 2 et 3.

nous le savons tous, l'ADN de la France est étroitement lié aux espaces ruraux et à la ruralité, tant sur le plan de sa géographie que de son histoire. La ruralité, ce sont de nombreuses petites communes qui présentent des situations très diverses, mais qui doivent toutes faire face à de nouveaux défis pour maintenir leur population et surtout leur activité économique. La revitalisation des centres-bourgs est un sujet fondamental sur lequel la puissance publique doit se pencher plus que jamais aujourd'hui, comme le Sénat l'a récemment fait pour enrayer la désertification des territoires ruraux. Cela doit passer par de nombreuses actions : faire disparaître les zones blanches en assurant l'égalité numérique de tous les territoires, maintenir et développer les réseaux de transport en commun, lutter contre les déserts médicaux en développant les maisons de santé pluridisciplinaires, préserver les dotations des communes rurales pour leur permettre d'investir dans des projets structurants, maintenir des services publics ouverts pour répondre aux demandes des usagers, inciter les entreprises et les artisans à s'installer dans les zones rurales. Lutter contre la désertification des territoires ruraux passe aussi par le maintien de commerces de proximité, véritables acteurs du maillage territorial et du dynamisme de la ruralité. Pour les préserver, des politiques publiques incitatives peuvent et doivent être mises en place. La lutte contre la désertification bancaire en fait partie. En effet, la disparition des agences bancaires en zone rurale marque l'accélération de cette désertification. Cette tendance trouve sa source à la croisée de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, nombreux sont les clients qui fréquentent de moins en moins leur agence, notamment avec le développement des services en ligne. Or le déplacement qu'un client est prêt à effectuer est d'autant plus long que ses besoins sont importants.

Dans ce contexte, les agences bancaires font le choix de se recentrer sur les zones urbaines, puisqu'elles considèrent que la proximité géographique n'est plus nécessaire. Clairement, les petites villes sont directement affectées par les conséquences du phénomène de raréfaction, voire de disparition des distributeurs automatiques de billets. estime que, entre 2008 et 2014, la France a perdu plus de 1 100 agences, soit une diminution de 2,8 % de son parc. Notre pays est passé sous la barre des 37 000 agences en 2016. Sia Partners prévoit que les banques passeront même à 34 000 agences en 2020.

Les banques mutualistes ont une emprise locale forte et garantissent une proximité avec leurs clients locaux et les pouvoirs publics. Cette présence est un avantage contre la désertification et le redimensionnement bancaires. En effet, il est difficile de fermer des agences dans une commune lorsque ces banques

La Banque postale porte une part importante des coûts du réseau des bureaux de poste. Elle compte plus de 17 000 points de vente, soit le double de ceux des banques LCL, Société générale et BNP Paribas réunies. Une réduction du maillage de cette banque aurait donc un effet très significatif sur le nombre total d'agences en France. Nombre de communes se trouvent confrontées à cette situation, qui suscite beaucoup d'incompréhension. Une fois encore, les élus locaux sont sollicités pour tenter de résoudre des problèmes qui ne sont pas de leur ressort, mais qui ont un fort impact sur la vitalité des centres-bourgs. À l'heure où les usages automobiles sont remis en cause,

S'il existe aujourd'hui des alternatives aux DAB, ... Il faut conclure, mon cher collègue ! ... comme la technique du ou du paiement sans contact, celles-ci représentent un investissement que tous les petits commerces ne peuvent pas se permettre. Une directive européenne sur les services de paiement est d'ailleurs entrée en vigueur cette année, mais demeure encore peu pratiquée.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, 92 % des Français plébiscitent aujourd'hui la carte bancaire pour leurs achats quotidiens.

La proposition de loi que nous examinons entend pérenniser la présence de distributeurs automatiques de billets dans les communes victimes de désertification bancaire. d'une désertification qui se traduit souvent, comme l'explique d'ailleurs le texte de nos collègues, par une baisse du chiffre d'affaires des commerces locaux, voire une fermeture de ces commerces au profit des grandes surfaces en périphérie et du commerce sur internet. Si nous partageons ce constat, nous divergeons sur les moyens à mettre en oeuvre pour répondre à cette question. Il aurait été opportun, me semble-t-il, que cette proposition de loi soit plus précise sur les différentes causes à l'origine de la diminution du nombre de DAB dans l'Hexagone ainsi, d'ailleurs, que dans le reste de la zone euro. J'ai déjà évoqué la diminution du nombre des retraits bancaires. Je pourrais aussi parler de la digitalisation de l'activité bancaire sur internet et des applications mobiles. L'usage croissant de la carte bancaire rend également les pièces et les billets plus rares dans les porte-monnaie, surtout depuis l'arrivée du paiement sans contact et de l'abaissement progressif du seuil d'acceptation de la carte bancaire par les commerçants, qui est désormais de 1 euro. En outre, les banques proposent ou expérimentent désormais des partenariats avec des magasins pour permettre à leurs clients d'avoir accès au sans avoir besoin d'un automate. exemple le Compte-Nickel, proposé par 3 800 buralistes, ou encore le, service de retrait d'argent liquide à la caisse des magasins, légalisé en France depuis la loi du 3 août dernier. En définitive, il ressort de ces observations que les moyens de paiement sont plus diversifiés que par le passé et ne reposent plus uniquement sur le réseau bancaire. Il n'en demeure pas moins que l'utilisation des espèces demeure essentielle, en particulier pour certaines transactions quotidiennes et de proximité. Ajoutons que les nouveaux usages ne concernent pas l'ensemble de la population : pour certains de nos concitoyens peu familiers des usages digitaux, le recours aux espèces reste vital. Quelles solutions peut-on dès lors envisager pour garantir la délivrance d'espèces sur tout le territoire ? Plutôt que de subventionner les communes pour qu'elles conservent ou créent leurs DAB, comme le suggèrent les auteurs de cette proposition de loi, nous soutenons la proposition de la rapporteur Sylvie Vermeillet visant à financer par le FISAC, dont le Sénat propose le rétablissement des crédits, l'installation de DAB dans les commerces de proximité situés dans les communes non couvertes par un réseau de radiocommunication mobile. Dans ces communes, les terminaux de paiement par carte bancaire ne peuvent pas fonctionner correctement, ce qui exclut le recours au, d'où l'importance de prévoir un accès aux espèces pour les habitants qui y vivent. L'instauration d'un critère de distance minimale des bureaux de La Poste comportant un DAB, prévue à 2, nous semble compliquée à mettre en oeuvre, car elle soulève d'importantes difficultés techniques, pratiques, juridiques, voire des difficultés en termes de sécurité. D'abord, La Poste assure déjà un service de mise à disposition d'espèces dans ses différents points de contact, qui suffisent à couvrir les besoins quotidiens. Ensuite, une extension de la mission d'aménagement du territoire assurée par La Poste nécessiterait de prévoir une compensation complémentaire, soumise au cadre européen relatif aux aides d'État, dont le principe actuel a été validé en avril dernier par la Commission européenne, et ce jusqu'en 2022. Compléter cette mission reviendrait donc à ouvrir la boîte de Pandore et à remettre en cause la sécurisation juridique de cette compensation. Enfin, cette compensation consiste en un allégement de fiscalité locale, non compensé par l'État. Le dispositif proposé serait donc supporté par les collectivités territoriales, alors que celles-ci ont déjà du mal à faire face à leurs obligations en raison du désengagement financier de l'État.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux est un objectif que nous partageons tous dans cet hémicycle. Aujourd'hui, quel est le constat ? Éric Gold et les membres du groupe du RDSE déplorent- à juste titre -les multiples fermetures de distributeurs automatiques de billets en zone rurale.

pour les résidents de ces zones, ainsi que pour les communes désertées en tant que telles, avec les conséquences que l'on connaît pour leur attractivité. Aujourd'hui, le contexte dans lequel s'inscrit cette problématique est bien celui d'une révolution des usages bancaires, avec l'essor de nouvelles technologies un recours plus fréquent à la carte pour des achats directs, comme le paiement sans contact. C'est pourquoi ce phénomène dépasse largement nos frontières.

En Franconie, région située au nord de la Bavière, la a lancé en 2015 un concept d'agence itinérante, afin de maintenir un service de proximité. Il est clair que les équipements bancaires, quels qu'ils soient, leur présence même ou leur maintien en état de bon fonctionnement participent de la vitalité économique des centres-bourgs. Cette question nous anime évidemment et continûment ici au Sénat, car cette désertification Une partie des usagers fera le choix d'une consommation extérieure à leur lieu de résidence, et ce pour des consommations courantes qui auraient pu rester locales. Ce sont les grandes surfaces en périphérie et en entrée de ville qui en bénéficieront alors, ou les acteurs du e-commerce. Autre risque : une partie des clients, ceux-là mêmes pour lesquels les déplacements sont rendus difficiles ou impossibles du fait de leur âge, par exemple, se sentiront légitimement marginalisés en raison d'un accès limité à ce type de service. C'est pourquoi le texte que vous défendez aujourd'hui dans l'hémicycle vise à maintenir ou à créer ces distributeurs dans les communes qui souffrent de ce que vous appelez la « désertification bancaire Afin de renforcer le maillage territorial des bureaux postaux avec les DAB, il est envisagé de créer un fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations, ciblé sur les territoires les plus en difficulté, c'est-à-dire les territoires dont les populations sont peu

Derrière ce dispositif se pose la question, qui ne se limite pas aux DAB, du recours aux espèces et de leur disponibilité. Alors que l'utilisation de la monnaie demeure encore essentielle, ce texte nous donne l'occasion de débattre- et c'est important -des conditions d'accès aux espèces,

Celle-ci est désormais prévue par le code monétaire et financier. Il faudra mesurer l'impact de cette mesure dans les territoires les moins bien pourvus.

risque existe d'un désengagement des opérateurs privés du maillage territorial en distributeurs automatiques de billets. Cette substitution doit rester l'exception. Le comité de pilotage de la filière fiduciaire, animé par la Banque de France, a mandaté un groupe de travail sur l'accessibilité aux espèces. Celui-ci devrait rendre ses conclusions d'ici peu, notamment sur la détermination des territoires les plus affectés par ces difficultés. Ce constat exhaustif et fiable des situations de défaillance avérée dans l'accès aux espèces sera important, afin de déterminer les critères géographiques, démographiques ou économiques,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Évidemment, le débat qui nous occupe aujourd'hui présente un lien assez étroit avec les préoccupations exprimées par nombre de nos collègues élus locaux à l'occasion de ce congrès. Le sujet qui nous intéresse est pour le moins important. Une partie de la France doit-elle, dans les faits, être privée d'entrer dans le XXIsiècle ? Les établissements de crédit agréés n'ont-ils pas quelques missions de service public et d'aménagement du territoire à accomplir ? L'accessibilité bancaire est-elle un mythe et un rêve quasi inaccessible ? ? Ces questions sont au coeur de la proposition de loi déposée par notre collègue Éric Gold, que nous ne pouvons évidemment que soutenir par principe, et qui mérite analyse. Ce que soulignent les auteurs de ce texte, et qui dépasse largement la question de la présence physique des distributeurs automatiques de billets de banque, c'est qu'une large qu'une large partie du territoire national n'est, encore une fois, pas placée dans les meilleures conditions pour participer à la vie sociale et économique du pays. Cette France rurale, « périphérique » dit-on aujourd'hui, de moins en moins tournée vers l'agriculture et de plus en plus transformée en villégiature pour ménages de salariés des grandes agglomérations, nous la connaissons tous très bien. Je suis moi-même élu d'une petite commune du Nord, dont la population a pourtant crû de près d'un tiers en vingt ans. J'ai été confronté, comme beaucoup d'entre vous, au refus obstiné des établissements financiers, à commencer par La Poste, d'améliorer leur qualité de service dans ma commune. Celle-ci se situe pourtant dans le périmètre de la métropole européenne de Lille. Notre collègue Éric Gold, dans sa communauté de communes proche de Clermont-Ferrand, sait très bien lui aussi ce que signifie cette lente et sûre progression de sa population.

Nous ne pouvons accepter une telle situation dans notre République, car elle met en cause l'égalité entre les territoires, lesquels sont les victimes d'une version abrupte de la concurrence libre et non faussée qui exclut ainsi, peu à peu, les lieux et les habitants de la périphérie pour ne s'intéresser qu'aux positions centrales.

la Cour des comptes selon laquelle « la question de la disponibilité des services bancaires sur le territoire et de l'inégal accès à ces services doit être examinée au regard de la diminution des services de guichet. [ ...] Seule La Banque postale, en raison des contraintes de présence territoriale imposées à La Poste, fait figure d'exception La Banque postale, justement : cela fait quelque temps que La Poste est, de manière historique, l'opérateur de référence pour l'accessibilité bancaire, tenu de permettre à toute personne qui le souhaite d'ouvrir un compte d'épargne ou un compte chèque. En foi de quoi, sur présentation du compte retraçant ces obligations de service public, La Poste se trouve ainsi rémunérée. Mais les banques ordinaires dans tout cela ? N'ont-elles aucune obligation

sur table. Côté face, nous devons prendre en compte certaines réalités, qu'on le veuille ou non : les distributeurs automatiques sont de moins en moins utilisés par nos concitoyens. Confrontés à l'utilisation massive des cartes bancaires, les distributeurs automatiques ne font plus autant recette. Selon le groupement d'intérêt économique des cartes bancaires, il y aurait 68 millions de cartes bancaires en circulation en France en 2017, à l'origine de 564 milliards d'euros de transactions, ce qui souligne l'attractivité de ce mode de paiement Côté pile, le paiement en espèce ne perd pas pour autant la face ! Selon l'étude de la Banque centrale européenne publiée en novembre 2017, les espèces restent le type de paiement le plus populaire chez les commerçants, qui n'ont, d'ailleurs, pas d'autres choix que de les accepter. Elles représentent 79 % du nombre total des achats réalisés en magasin et 54 % de la valeur de ces paiements. Bien qu'exprimant une préférence pour les paiements par carte, les Français réalisent deux tiers de leurs transactions en magasin en espèces. Il s'agit principalement d'achats d'un faible montant, ce qui confirme le rôle des espèces, en France, dans le règlement des petits achats du quotidien. Or, face à la digitalisation du secteur bancaire, avec l'essor des comptes et des services en ligne, l'utilisation des téléphones portables pour effectuer des paiements, les banques sont de plus en plus nombreuses à procéder à la fermeture d'agences et, par conséquent, de distributeurs automatiques, rendant ainsi difficile l'accès aux espèces, moyen de paiement préféré des consommateurs français. C'est, d'ailleurs, C'est, d'ailleurs, sous l'angle de l'accès aux espèces que cette proposition de loi rédigée par notre collègue Éric Gold aborde la question de la désertification bancaire. Si l'ensemble du territoire est impacté par ces fermetures successives de distributeurs automatiques, il existe d'importantes inégalités entre le monde rural et les grandes villes. Il y a une surdensification dans les métropoles régionales ou, encore, à Paris. On constate ainsi un déséquilibre de l'offre bancaire, qui touche en priorité les personnes les moins riches, les aînés et le monde rural. À titre d'exemple, dans la Nièvre, dans la Nièvre, les migrations contribuent à accentuer le vieillissement structurel du département : les seniors sont plus nombreux à s'installer qu'à partir, et inversement pour les jeunes. Ce Ce département, tout comme les autres territoires ruraux, doit faire face à des populations de plus en plus vieillissantes. Même si ces dernières ne sont pas nécessairement réticentes à l'évolution des modalités de paiement, des habitudes se sont créées, et une part importante de la population a besoin d'espèces. Les habitants des campagnes, des bourgs et des petites villes ont aujourd'hui ont aujourd'hui accès à un nombre toujours plus faible de distributeurs automatiques de billets. Cela les oblige à parcourir plusieurs kilomètres pour retirer de l'argent. Ils peuvent également se trouver confrontés à l'hostilité des commerçants, qui refusent parfois la carte bancaire pour des raisons économiques liées au coût du matériel et aux commissions prélevées. Face à cette désertification bancaire, des initiatives existent et ont été renforcées- elles ont été rappelées par de précédents orateurs. Nous avons par exemple ratifié, en juillet dernier, la directive européenne sur les services de paiement, qui concerne le. Dans les zones rurales, particulièrement, lorsque l'accès aux espèces est de plus en plus compliqué, le commerçant a la possibilité de distribuer manuellement des espèces. Ces opérations permettent, d'une part, de remettre les espèces au coeur de la stratégie des petits commerçants, en tissant du lien social entre les consommateurs et les commerçants, et, d'autre part, de redynamiser le commerce de proximité, ainsi que les centres-villes. Cependant, le n'est qu'une solution pour lutter contre l'absence de distributeur ; il ne peut combler le manque à lui tout seul. Les distributeurs automatiques sont indispensables aux petites communes rurales. C'est un service à la population qui participe à la sauvegarde du commerce local, pour lequel tous les élus se mobilisent chaque jour. Il s'agit là d'un enjeu lié à l'aménagement du territoire, comme on l'évoque régulièrement au sein de cette assemblée. Récemment encore, nous avons adopté à l'unanimité la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs de nos collègues Martial Bourquin et Rémy Pointereau. Les Français eux-mêmes sont inquiets de ce déclin des centres-villes. Une enquête réalisée par l'institut CSA, en juin dernier, auprès d'un millier de Français, montre que sept Français sur sont préoccupés par cette désertification. Nos coeurs de ville et de bourg meurent ; plus de 700 villes se trouvent en grande difficulté, tout comme plusieurs centaines de bourgs, pôles de centralité. Le plan gouvernemental « Action coeur de ville », lancé en mars 2018, est une première étape, qui permettra à quelque 200 villes de bénéficier d'une convention de revitalisation de leur centre. Mais le chemin est encore long pour redonner de l'attractivité à nos départements ruraux. Les maires et, plus largement, les élus locaux peinent à maintenir la présence des services publics, ainsi que des commerces de proximité. Beaucoup vous diront même que conserver un distributeur automatique de billets en milieu rural s'apparente, parfois, à un combat de haute lutte en termes de négociation avec les établissements bancaires. Cette question soulève- vous l'aurez compris, mes chers collègues -d'autres problématiques, très prégnantes dans nos territoires ruraux. La ruralité n'est en rien hostile aux évolutions numériques. Bien au contraire, elle réclame des infrastructures, des réseaux pour se connecter au reste de la France et au monde Les habitants qui la composent ne sont pas plus exigeants que les autres. Ils ne demandent qu'à avoir un égal accès aux services minimums présents dans les métropoles et les grandes villes ! Pour ces raisons, le groupe socialiste et républicain a accueilli avec beaucoup d'intérêt la proposition de loi de notre collègue Éric Gold. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen a souhaité que nous débattions, ce jour, de la proposition de loi de notre collègue Éric Gold, car elle tend à répondre à l'un des nombreux aspects de la relégation affectant nos territoires ruraux. En soutien aux élus locaux, le législateur doit veiller à préserver nos campagnes d'une désertification croissante, qui contribue à alimenter le cercle infernal de l'isolement. Cette désertification, nous ne saurions l'accepter, telle une fatalité ! Nous ne nous y résignons pas, soucieux de l'égalité entre tous les Français, attentifs à l'équilibre du territoire national et respectueux de la diversité qui fait la richesse et l'attractivité de notre pays Cette approche du monde rural, si elle est familière à notre Haute Assemblée, ne l'est pas nécessairement à toutes les sphères de pouvoir ou à celles et ceux qui les inspirent.

à cesser d'investir massivement dans une impossible égalité des territoires et à assumer que les territoires éloignés des grandes métropoles vont en partie être oubliés. Quel aveuglement sur le rôle que continuent de jouer ces territoires, en dépit de leurs difficultés, dans la dynamique nationale ! L'une de ces difficultés revêt aujourd'hui la forme d'une raréfaction des distributeurs automatiques de billets, elle-même s'inscrivant dans une tendance générale de raréfaction du recours aux espèces. Toutefois, les mutations des usages bancaires que nous observons, tout comme les évolutions juridiques tendant à réduire la capacité de paiement en espèces, ne sauraient masquer une autre réalité celle d'une partie de la population encore très peu en phase avec ces nouveaux usages, mais également celle de territoires ne disposant pas d'une couverture numérique permettant le recours à ces pratiques ou encore celle de commerces dont l'activité modeste en milieu rural tend à limiter le recours aux paiements dématérialisés pour des questions de coût. Aussi, la présente proposition de loi tend à faciliter l'accès aux espèces, en favorisant la présence de distributeurs automatiques de billets au sein des territoires,

cette problématique est très significative ; la Banque de France a d'ailleurs mandaté un groupe de travail sur le sujet. Sans préjuger aucunement de la qualité des travaux conduits par ce dernier, le groupe du RDSE a estimé qu'il était dans son rôle, en étant aussi force de propositions sur le sujet. Nous proposons donc la création d'un fonds dédié. Il nous est apparu

dont les derniers contours doivent être prochainement fixés, nous savons que ces dispositifs ne sont pas en mesure de pallier totalement l'absence de distributeurs automatiques de billets. de billets. Les usagers demeurent notamment contraints par les horaires d'ouverture des commerces proposant ce type de services. Mes chers collègues, la révolution monétique est engagée. Comme toutes les mutations, elle s'accompagne d'une période transitoire. Veillons à ce que celle-ci soit conduite avec réalisme et cohérence ! Aujourd'hui, on observe aisément que ce sont d'abord les populations urbaines qui réduisent leur recours aux espèces. Dans le même temps, ce sont les populations rurales qui souffrent le plus de la raréfaction des distributeurs automatiques de billets. La dématérialisation progressive des paiements est une composante que personne ne contestera ici. Toutefois, les premières pièces de monnaie ont été frappées au VII siècle avant notre ère ... Il me semble que nous pouvons nous employer à accompagner les usages propres à chaque territoire

La ruralité a besoin de proximité dans l'offre de services, au moment où le renchérissement du coût des déplacements dans ces territoires fait débat. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à nous accompagner et à nous soutenir, sans attendre la conclusion des travaux du groupe de travail mandaté par la Banque de France,

ruralité, à l'enjeu de l'écologie et de la protection de la biodiversité, qui doit être au coeur de nos politiques publiques ? Peut-on répondre, sans l'agriculteur

Pour en revenir plus précisément à la question de la désertification bancaire et de la raréfaction des distributeurs automatiques de billets et du paiement en espèces, il faut être lucide ! Comme plusieurs orateurs l'ont on ne peut pas envisager l'avenir en s'arc-boutant sur des schémas du passé ! Nier la réalité est toujours garantie de contre-performance ! La nature des services évolue bien chaque jour, et elle évoluera encore le numérique transforme notre société et, demain, cette transformation numérique emportera sur son chemin, et les paiements en espèces, et, je le crois, les paiements par chèque. Il est de notre responsabilité de regarder cette réalité en face. Nous devons nous y préparer.

conclusion, nous pensons, au sein du groupe de l'Union Centriste, que tant que le paiement en espèces existe, il faut maintenir un réseau de distributeurs automatiques de billets de proximité dans la ruralité. Nous sommes donc

Hier, on supprimait les agences bancaires ; aujourd'hui, les distributeurs. Au-delà de la seule suppression de ces distributeurs, c'est le processus dans lequel nous sommes entrés qu'il convient d'arrêter Plusieurs de nos collègues du groupe du RDSE, au premier rang desquels Éric Gold, nous soumettent cette proposition de loi visant à favoriser le maintien ou la création de distributeurs automatiques de billets dans les communes victimes de désertification bancaire. Ce texte a le mérite de soulever de vrais problèmes et d'amorcer un débat qui entre parfaitement dans le cadre du combat actuellement mené par le Sénat en faveur des territoires. Il faudrait, en effet, être aveugle pour ne pas constater cette diminution

Actuellement, nous constatons que les banques incitent de plus en plus à diminuer les échanges bancaires avec de l'argent numéraire, pour accroître l'utilisation des cartes bancaires, avec ou sans contact. Ainsi, elles réduisent les frais de fonctionnement liés aux transports de fonds, la maintenance des distributeurs automatiques de billets, et peuvent constater une augmentation des échanges, puisqu'il est plus facile de dépenser avec une carte qu'avec de l'argent numéraire. Mais cette évolution ne profite pas qu'aux banques ! Pour l'État, c'est plus de transparence sur tous les échanges financiers, donc moins de travail dissimulé.

Il est donc primordial de garder les points bancaires dans toutes les zones, pour maintenir les commerces de proximité et les TPE. Pour autant, faut-il une loi spécifique pour les banques ? À titre personnel, j'avais accueilli cette proposition de loi avec un positif, mais, au fil de la lecture du texte, je suis resté sur ma faim. J'ai été étonné de trouver si peu de chiffres, sur le nombre de distributeurs ou les échanges interbancaires, alors même que ces éléments servent de fondement à l'exposé des motifs. L'article 1, traitant de l'instauration d'un fonds dédié au maintien et à la création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales,

Les établissements de crédit, dans notre pays, sont soumis au contrôle et à l'agrément d'exercice délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui constituent une qui constituent une sorte de passeport fort utile pour la représentation de l'établissement auprès des instances officielles, pour faire jouer, le moment venu et au cas où, la solidarité de place. Leur contribution au fonctionnement de l'ACPR- aujourd'hui plafonnée, soit dit en passant -pourrait d'ailleurs se trouver quelque peu majorée, dans des proportions infimes, pour permettre à l'autorité de mener toute investigation nécessaire à l'appréciation de la « qualité de service » offerte aux usagers de tel ou tel réseau. cet amendement, nous proposons que l'agrément de l'ACPR porte aussi sur le projet stratégique d'implantation de l'établissement. Régulièrement, celle-ci examine les efforts accomplis par les réseaux bancaires pour être au plus proche des des usagers bancaires, notamment parce que la diversité des enseignes et des services proposés au public est la raison d'être d'une qualité de services financiers, telle que nous pouvons aujourd'hui la concevoir, et que cela n'est sans doute qu'un moindre mal au regard de la qualité de la « protection mutuelle » accordée par l'ACPR aux établissements de crédit dans leur ensemble. Quel

je comprends l'objectif de votre amendement, qui est d'assurer un recensement régulier des conditions d'accès aux services bancaires sur le territoire. Cependant, il ne me semble pas viser l'organisme pertinent, puisque ces missions relèvent de la Banque de France, dans une vision transversale à l'ensemble des établissements bancaires. C'est d'ailleurs sous son égide que les travaux du groupe de travail sur l'accessibilité aux espèces sont conduits. Les conditions de délivrance de l'agrément bancaire prévues à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier concernent des critères prudentiels, l'exigence de capital minimum par exemple. L'ACPR est compétente également pour assurer la protection du consommateur face aux pratiques commerciales déloyales, ce qui ne relève pas du champ visé par cet amendement. Je vous suggère donc de retirer votre amendement,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, les difficultés qui viennent d'être évoquées par nos collègues à l'instant sont bien réelles. La perte d'un DAB sur un territoire, en particulier en zone rurale, est véritablement une petite catastrophe. Et chacun sait ce que cela signifie pour nos communes lorsque ce service de base disparaît inévitablement, cela s'accompagne d'une baisse du chiffre d'affaires pour les commerces locaux, parfois de la fermeture de ces commerces au profit des grandes surfaces en périphérie et du commerce sur internet. Nous avons véritablement besoin d'un maillage territorial de bureaux de poste avec DAB sur nos territoires et il faut permettre aux communes d'être subventionnées afin soit de conserver le dernier distributeur, soit d'en créer un dès lors qu'il ne s'agit pas d'un distributeur automatique de billets associé au réseau de La Poste.

Tant la diminution du nombre de retraits que la digitalisation de l'activité bancaire, dont vous avez évoqué l'usage croissant, ou le développement de points de délivrance d'espèces autres que les DAB, que vous avez mis en avant pour choisir de ne rien changer, ne constituent de raisons valables pour justifier votre rejet

L'État n'a pas vocation à compenser les défaillances des banques sur le territoire ; il me semble donc plus approprié de s'appuyer sur la contribution de celles-ci dans une logique de responsabilisation sociale et territoriale. Le fonds de maintien et de création de DAB est un outil à la main de maires, dont la souplesse s'adapterait à chaque territoire. Une initiative locale présiderait toujours au déclenchement du fonds et à l'évaluation du montant de l'aide, et l'intervention dans le temps se ferait en fonction des situations locales, sous l'administration que le financement de ce fonds vienne limiter l'aide apportée aux collectivités dans d'autres domaines, puisqu'un gage permet de compenser les conséquences financières de sa création. L'option de l'extension des missions du FISAC pour aider les commerçants à implanter ces DAB, et ce uniquement dans les zones blanches, ne peut pas convenir, surtout dans le cas très probable du maintien du FISAC en gestion extinctive en 2019. Cela fait peser encore une fois sur le budget de l'État et sur l'initiative d'acteurs privés non rémunérés le maintien d'un service bancaire. C'est la même logique que celle qui mise sur le, qui représente un coût dissuasif pour les commerçants. Par ailleurs, ces deux options laissent les territoires dépendants des horaires d'ouverture limités des commerces locaux, ce qui est dommageable pour le dynamisme local. Je pense que, même dans les zones bien couvertes par le réseau numérique, où le peut trouver à s'appliquer, il faudrait proposer aux territoires un accompagnement de transition. Le conditionnement de la prime du fonds d'épargne à la qualité de l'implantation territoriale serait une incitation insuffisante, à mon avis, pour engager les banques à se déployer davantage sur les territoires. Je souhaite, avant toute chose, qu'une solution soit trouvée pour les territoires victimes de désertification bancaire. Ma préférence se porte évidemment sur un fonds interbancaire,

l'article. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais réagir à mon tour à la réponse du Gouvernement au phénomène de désertification bancaire. Si j'ai bien compris, il mise tout sur l'organisation programmée pour le début de 2019 du service de, dont on attend les décrets d'application. Cette solution unique ne prend pas en compte le fait que, dans les territoires les plus reculés, le réseau téléphonique et le réseau internet alimentant les terminaux de paiement par carte sont parfois très faibles, empêchant alors toute continuité de paiement. Cette alternative me semble non opérationnelle dans les zones à la fois non couvertes par le réseau internet et désertées par les banques. Toutefois, même dans les zones bien couvertes par les réseaux, il me semble que l'application du dès la fin de 2018 n'assurera pas un accès rapide aux espèces pour tout le monde. Son coût dissuasif pour les commerçants- d'ailleurs, pourquoi ne seraient-ils pas rémunérés pour assurer ce service bancaire -, la limitation de l'accès au liquide aux horaires d'ouverture des commerces, ainsi que la démographie vieillissante des territoires les plus désertés, qui ont des habitudes de paiement en liquide, en sont la preuve. La proposition de Mme la rapporteur se limite aux zones blanches ; or je pense que l'on ne peut résoudre ce problème dans sa globalité sans une réponse à la main des maires, suffisamment souple pour prendre en compte les besoins des différents territoires. La parole

pression de l'opinion des électeurs, tandis que nous, sénateurs, sommes les porte-voix, les porte-parole des territoires, à la fois dans leur diversité, mais également dans leur capacité à construire. Le sujet que nous abordons cet après-midi révèle parfaitement le malaise de la France aujourd'hui.

minimums et indispensables pour pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, certains s'amusent à théoriser et à planifier la fin du numéraire dans notre pays. Tout d'abord, nous n'en sommes pas là. Est-ce d'ailleurs une bonne chose ? Je n'en suis pas si sûre. En tout état de cause, d'ici là, on ne peut pas exiger

Il importe donc d'assurer à ces territoires un accès effectif aux espèces en précisant que, parmi les opérations actuellement éligibles au soutien du FISAC, figure l'adaptation des commerces de proximité en vue d'assurer la délivrance d'espèces. Ces commerces doivent être soutenus en vue d'accueillir en leur sein un distributeur automatique de billets en tant qu'agents d'un établissement bancaire au sens de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de préciser expressément cette possibilité

les établissements de crédit ordinaires ont la possibilité de proposer à leur clientèle de détenir un livret A, à l'instar de ce que faisaient jusqu'alors les caisses d'épargne et La Poste. Dix ans plus tard, l'essentiel de la collecte du livret A et de son frère cadet, le livret de développement ce qui n'empêche pas les banques ordinaires d'en bénéficier également. Pour autant, les établissements de crédit banalisés, autorisés depuis 2008 à participer à la collecte du livret A, perçoivent une commission de rémunération sur les encours qu'ils sont amenés à gérer. Ladite rémunération est fixée à 0,4 % du montant de l'encours, ce qui, dans une période de forte incitation à l'épargne, peut finir par représenter une somme non négligeable- plusieurs centaines de millions d'euros -, dégageant quelques ressources pour justifier un effort d'implantation dans les parties les moins attractives de notre territoire du point de vue de la stricte rentabilité financière. cet amendement, nous proposons donc que les établissements quelque peu réticents quant à l'affirmation de leur présence sur le territoire soient amenés à subir une moindre rémunération des encours de leurs livrets d'épargne, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, tel que cela est précisé dans le code monétaire et financier. L'amendement

Comme vous le savez, le Gouvernement est très attentif aux difficultés d'accès au cash dans certains territoires- je l'ai déjà indiqué -et aux conséquences que cela peut avoir sur les habitants et le développement de l'économie locale. Cependant, la mesure inscrite dans la proposition de loi, qui ferait reposer sur La Poste et La Banque postale seules la responsabilité de l'accessibilité en tout point du territoire à un DAB, appelle de la part du Gouvernement des réserves, que j'ai rappelées dans mon propos introductif.

les zones blanches. Il dresserait ensuite un bilan des actions engagées par les pouvoirs publics pour améliorer l'accès aux moyens de paiement dans les territoires et par ses opérateurs, permettant d'envisager le cas échéant des initiatives complémentaires qui répondent à votre questionnement. Quel

J'insiste sur le besoin impérieux de l'abondement du FISAC, qui permettrait donc de réimplanter les distributeurs automatiques de billets là où il y en a besoin. Je précise que le FISAC permet de maintenir également 2 000 stations-service de proximité, d'innombrables commerces, et de soutenir aussi des artisans. Vous me permettrez donc d'insister sur ce besoin indispensable.

la Banque de France conduit actuellement elle-même un rapport en associant l'ensemble du monde bancaire et postal. Madame la secrétaire d'État, quelles que soient les conclusions de ce rapport, qui doit être remis au mois de janvier- votre rapport est prévu sous six mois

Par ailleurs, la Banque de France est déjà saisie de ce dossier, puisqu'un groupe de travail sur l'accessibilité des espèces, déjà à l'oeuvre, devrait rendre ses conclusions au début de l'année 2019.

secrétaire d'État, outre la question des délais et de cet amendement de dernière minute déposé par le Gouvernement, que, sur une proposition de loi d'initiative sénatoriale, le Gouvernement propose un amendement

et revenir sur ce que vous appelez les prestations alternatives. Tout à l'heure, j'ai regardé les résultats nets des banques. Vous nous avez expliqué le coût des DAB.

je me sens soit en, soit en décalage horaire. Or je ne fais que revenir de la porte de Versailles, qui est aujourd'hui la porte des territoires de France. J'ai entendu toute la matinée les maires s'exprimer sur leur volonté positive de porter leur territoire. Et je n'ose imaginer, madame la secrétaire les réactions qui auraient été les leurs- encore que je ne sache même pas s'ils auraient été capables d'une réaction -quand je vous entends proposer, avec beaucoup de sérieux, la rédaction d'un rapport. Je vous avoue sincèrement, madame la secrétaire d'État, avec beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de gravité, que, dans nos territoires, il est urgent aujourd'hui de maintenir de la vie, non seulement pour que les territoires ne meurent pas, mais pour que les gens cessent de se rebeller.

du territoire et de contractualisation avec les collectivités, à la fois sur les mobilités et les services. Dernier point, madame la secrétaire d'État, je vous avoue que je ne comprends pas,

car il est urgent d'agir et de donner des réponses.

et déjà les charges relatives à l'épargne qui est collectée sur les territoires, très largement supérieure aux encours d'emprunts contractés sur les territoires ruraux.

Ensuite, je rappellerai que de nombreuses études montrent à quel point les communes rurales, pourtant loin d'être aujourd'hui majoritaires en population, pèsent dans la dynamique économique du territoire national, preuve que rien n'est perdu, si l'on utilise les bons leviers. ont besoin tous les acteurs ruraux aujourd'hui ? D'un formidable coup de pouce à l'activité, de l'allégement des charges et de la fiscalité, de la simplification drastique des normes et des règlements qui étouffent les PME.

précisément de quels montants on parle, combien de DAB il faut installer, voire quelles sont les solutions alternatives, me semble correspondre à une façon assez raisonnable de travailler. Vous allez avoir du mal ! Je réponds à votre question sur le fait de rédiger un rapport plutôt que d'agir. Oui, nous agissons et nous avons agi beaucoup ces seize derniers mois, je suis heureuse que vous le souligniez. Mais il nous arrive d'agir en faisant un diagnostic, et c'est bien cela qui semble manquer aujourd'hui,

Commission européenne, du fonds qui finance ce dispositif, etc. Mon dernier point concerne les banques. S'il s'agit bien d'un service public, je crois me souvenir qu'il faut le compenser. Donc, c'est le contribuable qui devrait payer.

des gens des territoires. Ils manifestent, car ils se sentent oubliés. Or, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, il n'y a pas de « territoires reculés »- il est choquant d'entendre une expression comme celle-ci -, comme il n'y a pas de territoires « avancés

... La décision de transférer le bureau de poste à la mairie, avec une agence postale communale, permet aujourd'hui de donner à des retraités 300 euros par semaine, mais à condition d'avoir un compte à la Poste.

que cet amendement vise à mettre un point final à cette initiative et à ce texte, qui répond réellement à un besoin.

de la proposition de loi qui modifie la loi postale en y introduisant une norme supplémentaire d'accessibilité au réseau de distributeurs automatiques de billets de La Banque postale. Alors que cet article viendrait alourdir considérablement les obligations de La Poste en matière d'accessibilité, il n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. Or, du fait de sa mission d'aménagement du territoire, La Poste met déjà à disposition des clients de sa banque une large offre d'accès aux espèces. Ainsi, de septembre 2018, le réseau de La Poste comprenait 17 365 points de contact sur le territoire, dont plus de 8 000 bureaux de poste offrant l'offre bancaire complète, 6 300 agences postales communales et intercommunales offrant les services de retrait et de versement dans la limite de 350 euros par compte sur sept jours glissants, et près de 2 800 Relais Poste offrant les services de retrait et versement dans la limite de 150 euros par compte sur sept jours glissants. Bien entendu, une telle mesure représenterait une rupture d'égalité face à la loi. La proposition de loi propose la création d'un fonds de soutien, ainsi que des conventions avec les banques en général, pendant que l'article 2 fait peser uniquement sur La Poste la contrainte en termes d'accessibilité, en extrapolation des obligations de présence postale.

Toutefois, je tiens à rappeler que la digitalisation de ce secteur risque d'entraîner et d'accélérer les fermetures d'agences en France, et donc d'accentuer la désertification bancaire dans nos territoires ruraux. Aujourd'hui, 80 % à 90 % des souscriptions de produits bancaires sont réalisées dans les agences. Mais, dans deux ou trois ans, lorsque les banques auront achevé la digitalisation de leur parcours client, les volumes de souscription en agence vont radicalement baisser. cette évolution pour les personnes les plus éloignées du numérique, je vous propose d'obliger les établissements bancaires à informer le maire de la commune d'implantation avant tout projet de fermeture d'une agence, quant aux moyens mis en oeuvre pour garantir la continuité de l'accès à leur réseau.

J'approuve l'intention : il s'agit de ne pas pénaliser les commerçants et les consommateurs qui peuvent être contraints de recourir à la carte bancaire pour des transactions courantes. j'ai quelques doutes quant à l'application de ces dispositions. En pratique, les frais liés à l'usage de la carte bleue sont fixés dans une convention d'utilisation entre le commerçant et l'établissement bancaire. Comment les critères d'accès aux distributeurs automatiques de billets seraient-ils appréciés ? Comment les conventions seraient-elles justifiées ?

? Cet amendement vise à encourager l'acceptation de la carte bancaire par les commerçants dans les zones rurales où il n'y a pas de distributeur automatique de billets. rappeler que, sur l'initiative des pouvoirs publics et des autorités européennes, le montant des commissions à la charge des commerçants a été substantiellement réduit au cours des dernières années. La commission dite « interchange

sous l'égide du Comité national des paiements scripturaux, afin de faciliter l'acceptation des paiements par carte à partir d'une somme très faible. Les dispositions proposées risqueraient d'avoir des effets pervers : en définitive, elles iraient à l'encontre du but visé et pourraient rendre plus aigu le problème de desserte de ces territoires en modes de paiement adéquats.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons d'achever l'examen d'un texte à la fois pragmatique, en ce qu'il répond à un manque, et novateur, en ce qu'il propose un mécanisme inédit. À travers cette initiative transparaît notre ambition d'une meilleure cohésion des territoires. notre proposition de loi s'efforce d'apporter une réponse opérationnelle à une difficulté réelle rencontrée non seulement dans certains territoires ruraux, mais aussi dans certains quartiers de la politique de la ville

de répondre à ces attentes du quotidien. Le débat que nous avons choisi d'inscrire dans notre espace réservé a pu, par le passé, être abordé dans cet hémicycle. De plus, le Sénat, par son ADN, porte une attention particulière aux thématiques relevant de nos territoires, et notamment de nos zones rurales. D'autres le diront après moi : il n'existe évidemment pas un archétype de la ruralité. ruraux sont divers et s'inscrivent dans des dynamiques singulières. Notre débat vise également à sortir des caricatures et des postures. Oui, les gouvernements successifs ont mené des réformes. À cet égard, je salue le retour sur nos travées de Jacques Mézard. Nous connaissons tous la vigueur avec laquelle il a défendu, dans ses fonctions ministérielles, le développement de tous les territoires. Très bien ! Je pense non seulement aux villes moyennes, autour du plan national « Action coeur de ville », mais aussi aux zones rurales. Ces territoires, nous les connaissons, nous en venons, nous y retournons chaque semaine. Et je vois d'ailleurs que les orateurs qui me succéderont sont tous d'excellents connaisseurs des ruralités ! Monsieur le ministre, vous-même disposez d'une expertise certaine en la matière, puisque vous êtes ancien élu rural et chasseur.

vous m'avez souvent entendu tonner à cette tribune contre la limitation de la vitesse à quatre-vingts kilomètres par heure sur les routes nationales. Je note que cette mesure, dont je doute toujours de l'efficacité, contribue à allonger les trajets quotidiens de millions de personnes. Elle a aussi été perçue perçue comme une incompréhension des réalités vécues. En effet, pour beaucoup de Français, il n'existe pas, en tout cas pas encore, de moyen de se passer de la voiture individuelle. Cela explique sans aucun doute l'accès de fièvre qui touche actuellement notre pays, lequel voit nombre de nos compatriotes revêtir un gilet jaune. Monsieur le ministre, la question des mobilités est une dimension majeure de l'aménagement du territoire. Un projet de loi d'orientation, très attendu, devrait être prochainement inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres. Pouvez-vous nous éclairer quant aux dispositions qui s'appliqueront plus spécifiquement aux espaces ruraux ? Parmi les autres motifs de préoccupation, j'évoquerai tout d'abord l'accès à des soins de proximité et de qualité. En la matière, plusieurs actions ont été engagées ces dernières années, promotion de la création des maisons pluridisciplinaires ou le renforcement des mécanismes incitatifs à l'installation de médecins dans des zones sous-dotées. Nous avons évidemment porté une grande attention aux mesures du plan « Ma Santé 2022 », présenté en septembre la République. Ce plan ambitionne de réviser en profondeur l'organisation territoriale, pour la médecine de ville comme pour le maillage hospitalier. Sans entrer dans les détails, il s'agit de créer un collectif de soins de proximité à l'horizon de 2022.

Même si ces thématiques ne relèvent pas directement de vos attributions, pouvez-vous nous en dire davantage à propos de son impact sur la carte des hôpitaux de proximité ? L'accès aux services publics est une autre problématique récurrente. En la matière, les maisons de services au public, les fameuses MSAP, ont pu constituer une réponse intéressante en permettant de maintenir, des formes nouvelles, la présence de services au plus près de nos concitoyens. Comment entendez-vous poursuivre l'effort dans cette direction ?

publique, la MAP, succède aujourd'hui le plan Action publique 2022, qui suscite certaines inquiétudes. Le Gouvernement doit les entendre, surtout quand un même territoire est touché par des fermetures en cascade sans que les différents services de l'État semblent se concerter. souhaite également m'attarder sur la dimension numérique de l'aménagement. Nous le savons, l'accès à l'internet à très haut débit et la couverture mobile partout en France constituent un sujet de préoccupation majeure pour nos concitoyens. Alors que le numérique est présent chaque jour dans nos vies, l'accès à une connexion internet de qualité est devenu aussi important que l'accès à l'eau ou à l'électricité. Au regard des constantes innovations, nous sommes à l'aube de bouleversements plus grands encore, qui seront permis par ces technologies. Assurer leur développement partout et pour tous relève donc de l'égalité républicaine. Dans les espaces ruraux, le numérique peut constituer une formidable chance de dépasser certaines contraintes géographiques, à condition, bien sûr, que l'on dispose d'une couverture de qualité. C'est un défi considérable qui nous est collectivement posé, et pour lequel l'État, en partenariat avec les opérateurs de télécommunications et les collectivités territoriales, a décidé d'engager des moyens sans précédent, notamment dans le cadre du plan France très haut débit. ainsi une montée en puissance régulière, même si nos concitoyens trouvent que le mouvement ne va pas assez vite. Entendons leur impatience. Dans les zones peu denses, l'outil majeur est constitué par la mise en place de réseaux d'initiative publique, les RIP, qui bénéficient d'une enveloppe de subventions de l'État de 3,3 milliards d'euros. Les RIP se déploient dans les départements. Mais, ces derniers mois, s'est posée la question d'un nouvel abondement de l'État et de la réouverture du guichet de subventions.

pouvez-vous nous dresser un rapport d'étape, quant à la mise en oeuvre de l'accord historique de janvier dernier et quant à l'atteinte de l'objectif de généralisation d'une couverture mobile de qualité dès 2020 ? prégnants, ce qui commande de les inclure dans notre politique d'aménagement. C'est la raison pour laquelle nous avons milité, au début de ce mois de novembre, pour que l'Agence du numérique rejoigne la future agence nationale de la cohésion des territoires, dans le cadre de la proposition de loi que notre assemblée a adoptée.

ou le soutien à la vie culturelle. Mais, ayant évoqué les difficultés auxquelles font face les territoires ruraux, je ne voudrais pas alimenter le cliché d'une ruralité malheureuse. Si nous avons fait le choix d'inscrire ce débat à l'ordre c'est aussi pour mettre en avant les potentialités de ces territoires, et pour cause : il y a de la vie dans nos campagnes, il y a de l'espoir, il y a des initiatives qui fleurissent, et qui sont menées par des citoyens, des entrepreneurs ou des élus.

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de reprendre quelques chiffres clefs publiés par l'Association des maires ruraux de France 21,4 millions de personnes résident aujourd'hui dans une commune rurale, à savoir un Français sur trois ; 85 % de ces habitants sont des actifs potentiellement créateurs d'une activité économique compte 32 212 communes rurales, et plus de 80 % d'entre elles sont en croissance démographique. Contrairement aux idées reçues, la ruralité n'est pas nécessairement liée au monde agricole. Elle vit aussi grâce à des PME ou à de grands groupes. Les territoires ruraux sont une richesse en termes d'espace, de qualité de vie, de développement économique et de vie sociale. Le monde rural joue un rôle essentiel. Il présente un important potentiel de bâti à restaurer : nous pourrions y accueillir des locataires sans dévorer des terres agricoles et, ainsi, redynamiser les coeurs de village. Nous devons préserver le foncier agricole, même si l'agriculture n'est plus la composante unique de la ruralité. Avec l'accès à internet, les territoires deviendront attractifs. C'est une condition essentielle à la vie des communes. Pour le développement économique, la santé, l'école et la formation, le quotidien des habitants qui vivent en milieu rural, il est important de maintenir une véritable offre de services publics. Nous devons, ensemble, réaménager le service au public et en rendre l'accès facile à la population vieillissante. Les communes ont bien souvent investi pour réaménager des classes, construire des groupements pédagogiques et des cantines. Ces écoles sont des lieux de qualité. L'enfance y est belle. Il faut favoriser la desserte des villages afin que chacun puisse circuler correctement : les bus scolaires et les magasins ambulants sont autant de liens indispensables pour la population. Une bonne circulation routière, voire ferroviaire, avec la réouverture de petites lignes, favoriserait le développement économique. Peut-on donc encore légitimement parler d'une opposition entre urbain et rural ? Non, il faut apprendre dorénavant à échanger : l'équité s'impose, c'est la seule voie possible. Nous devons, enfin, voir la ruralité comme une chance pour notre pays, car elle est plus que vivante. Osons même dire qu'elle se mérite ! En septembre dernier, lors d'un congrès national des maires ruraux, j'ai perçu une profonde inquiétude chez les élus. eux se posent beaucoup de questions sur l'avenir et se sentent délaissés au profit des grandes agglomérations. Pourtant, malgré la diminution des compétences des maires, le monde rural avance et se développe. Les projets sont là, mais les dossiers pour obtenir des financements

pour faire sortir le pays de ses impasses, aidez-nous à nous occuper de nos populations, rendez-nous du pouvoir d'agir, donnez-nous un véritable statut d'élu qui accompagne l'engagement de ces centaines de milliers de bénévoles. » Quoi de plus beau, socialement, que la gestion d'une commune rurale ?

Aujourd'hui, le monde rural peut apporter beaucoup, à condition qu'il ne se sente pas délaissé ni injustement oublié. Il adresse ainsi un appel formidable aux investisseurs privés

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

la définition même du « rural », qui doit être plus précise, afin que l'on puisse mettre en place des actions spécifiques, efficaces, propres à chacun des territoires. Le périurbain n'est pas la campagne profonde. Il faut distinguer deux ruralités : la ruralité périurbaine et l'hyper-ruralité. La première La première est proche des villes et des centres d'emploi, elle est dynamique, elle attire notamment les jeunes couples et les retraités qui cherchent une qualité de vie entre ville et campagne, tout en maintenant la proximité des services publics, des activités culturelles et sportives. Dans ces zones, les maisons se vendent, les hameaux sont peuplés, le foncier se porte bien. Le développement de cette ruralité périurbaine est souhaité par les habitants pour la qualité de vie qu'ils y trouvent. C'est un atout fort de ces territoires, qu'il convient de soutenir davantage au travers de la mise en oeuvre de politiques publiques adaptées au niveau des communautés de communes et d'agglomération : aides au désenclavement, à la création d'emplois, programmes de voirie, développement des infrastructures et du numérique, préservation des services publics. Ces communes périurbaines

des territoires, avec une diminution constante de la population, comme dans les zones d'élevage, lesquelles ont connu un exode de leurs agriculteurs, dont le nombre a été divisé par quatre en

privées et attirer une nouvelle population. Cela est possible si la volonté existe ; malheureusement, depuis plusieurs années, tel n'est pas le cas.

en fonction de leur niveau d'enclavement, de leur densité de population, de leur distance par rapport aux axes autoroutiers et ferroviaires ou encore de l'éloignement des bassins d'emploi. Il faudrait également mettre en place un guichet unique sous l'autorité directe du préfet, qui centraliserait les dossiers de créateurs d'entreprises et d'initiatives publiques et les accompagnerait tout au long du processus de création, en bonne coordination avec les acteurs concernés du territoire : région, conseil départemental, agglomérations, communes et chambres consulaires. L'agence nationale de la cohésion des territoires, portée par Jean-Claude Requier, jouera-t-elle ce rôle ? Des avantages fiscaux et sociaux additionnels permettraient de compenser les inconvénients découlant de l'enclavement : des zones

Depuis trop longtemps, l'État ne considère pas l'hyper-ruralité comme une chance pour la France, mais plutôt comme des territoires sans avenir, des zones ignorées, en désertification.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, « La ruralité : une chance pour la France », voilà un beau sujet pour le grand oral de l'ENA, qui aurait ainsi l'occasion, pour une fois, d'évoquer cette autre France ! Bien entendu, ces territoires, peuplés par des autochtones d'un autre siècle, qui « fument des clopes et roulent au diesel », ont des atouts dans leurs mains ; à condition, toutefois, que l'État ne joue pas au poker menteur. C'est en partant de nos handicaps que nous trouverons les voies de notre développement. Cette volonté de partir des réalités pour imaginer l'avenir préside aux réflexions du groupe de travail consacré à la ruralité que j'anime avec mes collègues Daniel Laurent et Jean-Marc Boyer au sein du groupe Les Républicains du Sénat, Sénat, qui s'articulent autour de trois axes incontournables : le développement économique, les services au public et l'organisation territoriale. Elles s'inscrivent dans la continuité logique du précédent groupe de travail que j'avais eu l'honneur d'animer en 2016 et qui avait conduit à l'adoption de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural. Le Gouvernement n'a jamais jugé utile de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais le Sénat a obtenu des avancées en enrichissant la loi portant évolution du logement,

À quoi aspirent nos compatriotes qui vivent dans les bourgs et les villages ? À travailler au pays, à y disposer de services, notamment médicaux, et à habiter dans un logement qui corresponde à leurs besoins, leur culture et, surtout, leur façon de vivre. Avons-nous, depuis lors, beaucoup avancé sur ces attentes aussi légitimes qu'essentielles ? Comme beaucoup d'entre nous, j'en doute. Pour renforcer l'attractivité de nos territoires, qui offrent un cadre et une qualité de vie incomparables, la priorité reste l'emploi et donc le développement économique, qui nécessite un désenclavement routier, ferroviaire et numérique. Les citoyens, les entrepreneurs, les élus ruraux réclament moins de contraintes et de normes, mais davantage de marges de manoeuvre pour conduire des initiatives privées adaptées à leurs réalités. La proposition de loi sénatoriale portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs a été un premier pas important, mais il en faudra beaucoup d'autres pour réparer des décennies d'ouvertures d'hypermarchés aux conséquences ravageuses. commerce, le FISAC, que propose le Sénat dans le cadre du budget pour 2019, est une excellente chose, à condition de l'utiliser conformément à sa vocation : au profit des artisans et commerces de proximité. Pour créer ce nouveau souffle, il faut également une démographie plus dynamique, qui est indissociable du développement des services publics, évidemment, mais aussi des services à la personne, notamment dans le domaine médical.

L'organisation de notre République- décentralisée, paraît-il ! -est un levier important dans le combat pour la ruralité. Adaptons-la aux réalités géographiques, plutôt que l'inverse Dans le nouveau jardin à la française des intercommunalités « XXXL », il faut redonner aux communes les capacités d'agir, car elles sont l'échelon de base de la démocratie et font battre le coeur de nos territoires. Les premiers acteurs de cette vitalité que nous appelons de nos voeux sont les élus locaux. Monsieur le ministre, si, à l'occasion de la réforme des institutions, le nombre de sénateurs qui les représentent baisse jusqu'à devenir anecdotique, les régions rurales et leurs habitants, faute de défenseurs, sombreront définitivement dans l'oubli et le déni démocratique. Pour conclure, je rappelle que, pour tirer la France rurale vers le haut, nous demandons le soutien de l'État et non un discours de compassion porté par ses représentants. ses représentants. En 2015, 21 % de la population habitait dans une commune rurale de moins de 3 500 âmes ; il ne s'agit donc pas d'une frange marginale, mais d'un Français sur cinq. Les ruraux aiment et défendent les agriculteurs et l'environnement, mais ils veulent pouvoir tirer parti de leurs ressources sans vivre parqués dans des réserves à la population vieillissante et déclinante. Alors, réveillons nos territoires ! Offrons à nos concitoyens la possibilité d'exprimer le dynamisme dont ils sont capables ! Faisons confiance à leur aptitude à penser leur futur qui, loin de l'image figée du passé, projettera un avenir qu'ils auront eux-mêmes imaginé. Au nom des ruraux, je termine par un appel. Monsieur le Président de la République, mesdames, messieurs les ministres, cessez de nous ignorer et de nous mépriser, mais écoutez-nous, entendez-nous

toute leur place pour permettre le maintien de territoires dynamique, de territoires vivants, de territoires d'innovation, puisque l'innovation est une opportunité

Cette approche originale attire notre attention sur une spécificité française. En effet, poser la question de la ruralité, c'est s'intéresser à une somme de problématiques qui vont bien au-delà du portrait qu'on en faisait, il n'y a pas si longtemps encore, en désignant par ce vocable des territoires à l'activité majoritairement agricole.

Non, la ruralité ne peut pas faire seulement l'objet de discours condescendants ponctuels ou de quelques mesures destinées à compenser les carences dont elle souffre depuis plusieurs années et qui ne font que s'amplifier, alors qu'elle est riche de tant de potentiel, de talents, de créativité et d'énergies. Ces territoires sont d'abord des laboratoires de démocratie locale où la relation de proximité qui s'établit entre habitants et élus leur permet de débattre directement des choix et des projets.

les enseignants, toutes les forces vives qui garantissent une cohésion sociale rassurante et équilibrée. Personne ne reste sur le bord de la route dans ces espaces privilégiés de l'exercice de la démocratie. Ainsi, la création des services d'aide à la personne en milieu rural et leur développement témoignent de la capacité de ce système participatif à répondre aux besoins de tous ses membres. Ce n'est sans doute pas non plus par hasard que ces territoires sont également des laboratoires d'innovation qui génèrent des emplois dans des secteurs industriels nouveaux. Les visites d'entreprises que j'ai effectuées dans mon département, la Seine-Maritime, m'ont permis de découvrir, dans des communes d'où l'activité agricole a parfois presque entièrement disparu, des acteurs économiques travaillant dans des domaines très pointus et dont le rayonnement s'étend dans certains cas bien au-delà de nos frontières. L'espace rural devient alors un lieu de production de nouvelles richesses, tourné vers les énergies renouvelables en développant la filière bois ou la fabrication de plastiques ménagers à partir de matières recyclées

C'est précisément parce que notre territoire national dispose de ces richesses, qui lui confèrent son originalité, que nous devons leur permettre de s'exprimer et de prospérer,

retrait de l'État et de ses services, tel que les bureaux de poste ou les trésoreries, mais aussi fermeture de maternités, inégalités de desserte ferroviaire, désertification médicale, difficultés financières, disparition des petits commerces de proximité, distances toujours plus importantes à parcourir pour accéder aux services minimums. Alors que se tient le Congrès des maires, c'est l'écho de la désillusion des élus ruraux, pourtant si ambitieux pour leurs territoires, qui nous parvient.

Notre ruralité est belle, certes, et le nombre de touristes qui la parcourent chaque année confirme l'attrait qu'elle exerce et l'intérêt qu'elle suscite, mais elle ne saurait se contenter de devenir un musée à ciel ouvert Pour conclure, monsieur le ministre, nous ne cherchons pas à opposer le rural et l'urbain, mais nous rappelons que l'égalité des territoires est indispensable à l'équilibre du territoire national qu'il ne peut y avoir de sous-territoire comme il ne peut y avoir de sous-citoyen. La richesse est présente partout dans l'Hexagone, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue l'opportunité de ce débat, avant l'ouverture de l'examen du projet de loi de finances pour 2019. J'espère sincèrement qu'il sera possible d'adopter un changement de perspective et donc de politique publique à l'égard du monde rural. la ruralité constitue, selon l'expression du sociologue Jean Viard, une société vivante en passe de proposer son propre modèle de développement économique et social, qu'il faut impérativement identifier et accompagner.

des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières ». Or cette mesure n'a été ni mise en oeuvre ni même testée, alors que les élus de montagne Quelle est aujourd'hui la préoccupation principale des élus ruraux ? Ici, la préservation de l'école ou du collège, là, de l'institution publique, ailleurs, de la petite entreprise, partout, le combat permanent contre les mouvements de centralisation vers de trop grandes intercommunalités. trop grandes intercommunalités. En visitant les élus de mon département, je suis frappé par leur envie de construire un autre mode de développement, plus autonome, plus humain qui s'appuie sur nos ressources propres et qui s'inscrit dans une stratégie nationale d'innovation et d'expérimentation. Mes chers collègues, pour cela, nous avons besoin que des infrastructures minimales présentes dans tous les territoires. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous demandons ainsi depuis plusieurs années le désenclavement de la préfecture du département, Digne-les-Bains. Concernant la couverture mobile et le numérique, nous n'avons plus de temps à perdre au risque de voir partir des populations pourtant séduites par la vie rurale. Nous plaidons pour une couverture plus rapide, mieux priorisée, qui utilise les infrastructures existantes, comme les pylônes TDF, notamment, ainsi que les bornes 3G actuelles, qui pourraient être mobilisés maintenant, sans attendre une hypothétique 5G, partout où la fibre est déployée uniformément.

ainsi mettre en place un maillage plus cohérent de ces services au public. Les longues distances quotidiennes ne doivent plus être une fatalité pour la ruralité. Monsieur le ministre, nous avons besoin d'infrastructures adaptées. En retour, les élus ruraux sont prêts à agir en autonomie, à expérimenter et à innover. Il faut s'appuyer sur eux.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à chaque déplacement dans mon département de l'Aveyron, je ne cesse de répéter à tous mes concitoyens : « Soyez très fiers, vraiment très fiers, d'être des ruraux

pour alimenter et bâtir le pays. Bien sûr, il y a toujours eu des moqueries- nous nous les rappelons tous -sur les ruraux, qui ne seraient pas assez distingués, et l'exode rural est massif dans l'espoir de trouver un travail plus rémunérateur ailleurs. Néanmoins, la ruralité d'aujourd'hui n'est plus celle qui est fantasmée par les uns, dénigrée par les autres. Nous nous sommes développés, et la réalité est bien différente aujourd'hui nous aussi, nous disposons d'entreprises innovantes et performantes ; et, bien sûr, la qualité de la vie est, pour nous ruraux, bien supérieure- je le dis ici, à Paris -à ce qu'elle est dans d'autres endroits. En effet, nous avons un espace sain-

notamment celui de la jeunesse et du renouvellement des générations. En effet, nos départements ruraux vieillissent. Il nous appartient donc à tous de conserver toutes les qualités de notre territoire et d'attirer de nouvelles populations, surtout des entreprises qui créeront des emplois. il est nécessaire que les départements de moins de 300 000 habitants bénéficient d'actions spécifiques pour compenser leurs handicaps naturels

Pourquoi la majeure partie des collectivités locales- communes, communautés de communes et départements -de province ont-elles une dette plus élevée que les métropoles ?

Car c'est bien de l'attractivité qu'il s'agit. Alors que les métropoles et les départements urbains ne cessent de voir leur population progresser, le milieu rural, lui, se désertifie. Il est absolument impératif de rétablir cet équilibre. Les départements ruraux ne sont pas faits spécifiquement pour accueillir les touristes aux mois de juillet et août

territoire. Mes chers collègues, inventons un nouveau milieu rural : ainsi, certaines mesures ou certaines lois ne peuvent pas s'appliquer de la même manière à Paris et dans nos départements ruraux,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le concept de ruralité a toujours fait les délices des géographes et des parlementaires.

Et vous me demandez d'en parler comme d'une chance ? Vaste programme, au surplus dans un temps si bref que j'en frémis. Aujourd'hui, beaucoup définissent la ruralité par la négative, comme ce qui n'est pas la ville. Les travaux qu'elle inspire reposent sur une définition victimaire : la ruralité qui s'est conceptualisée est celle qui subit. Il est certain que la souffrance de nos campagnes est réelle, mais ce discours est-il une base saine pour défendre un projet de développement positif pour une ruralité du XXI siècle ? Alors que la ville a assis son rôle culturel, politique et économique, notamment dans son affirmation continuelle vers la métropole, la ruralité se cherche toujours un avenir dans notre époque. En d'autres termes, l'urbanité est un fait, quand la ruralité est un souhait. Il faut donc lui construire une vision et un projet pour qu'elle constitue une alternative. Elle doit cesser d'être une victime, bien sûr, mais aussi une utopie ou un objet désirable, pour devenir conquérante et se développer pour et par elle-même. Elle ne possède pas les mêmes atouts que la métropole, mais elle a les siens. Elle doit donc se donner la juste ambition de cesser d'être définie comme un legs du passé qui se contente de s'incarner dans le présent, pour devenir un projet d'avenir inscrit dans la modernité. modernité. Pourquoi miser sur ces territoires perdus et vouloir y vivre, malgré des dynamiques de développement plus faibles ? Parce que nos territoires sont davantage que des subjectiles dans le contexte de la rareté et de la préservation de notre environnement : ils sont un enjeu vital dans la guerre des ressources qui commence et doivent être vus, eux qui ont jadis bénéficié d'investissements lourds, mais parfois dépassés, comme les vecteurs du développement sur le temps long, en ces temps d'immédiateté. À cet égard, la ruralité du XXI siècle sera interconnectée ou ne sera pas. Le web 2.0, voire le 4.0, a révolutionné la géographie et les distances. S'il n'y a plus de ni d'Amérique à découvrir, les grands moments de développement se font ailleurs, et l'avenir des pionniers se situera toujours dans les marges abandonnées ou inexploitées. Le préalable incontournable est de renverser le paradigme de la fiscalité locale, locale, conceptualisée voilà plus d'un demi-siècle et fondée sur la territorialisation de la ressource et une affectation de celle-ci guidée par le nombre d'habitants. Cette approche, n'ayant plus aucune réalité contemporaine, constitue une véritable spirale du déclin, qui a vocation à fermer le spectre des dynamiques dans un conformisme réducteur et qui conduira à la sclérose de notre pays, si nous persistons. Mes chers collègues, la loi de finances exceptionnelle prévue au printemps prochain sera pour nous l'occasion de renouveler notre force créatrice et de saisir la chance à cet égard, pour peu que nous sortions de nos sempiternels lieux communs et de l'écosystème fiscal actuel, en osant appréhender les charges réelles et en refondant une nouvelle gouvernance systémique. Je vous y donne rendez-vous Si la cité semble avoir fondu son destin dans celui de la ville, nous proposons d'imaginer la cité rurale : elle n'est pas un destin, une voie tracée, mais un projet, un défi collectif de reconstruction des espaces et des usages, auquel il nous faudra retravailler. Ne nous trompons pas, la ruralité n'est ni vraiment une chance ni un boulet elle est l'avenir de notre pays, pour peu que nous souhaitions conserver ses valeurs, qui nous ont portés du premier sacre de Reims jusqu'à Charles de Gaulle, en passant par les Lumières et la Commune, des valeurs qu'une insidieuse société de consommation voudrait déconstruire. C'est la tâche que nous nous sommes fixée, à quelques-uns, en brûlant les images d'Épinal pour libérer la ruralité et élaborer ensuite des outils dans une architecture nouvelle permettant aux acteurs de se prendre en main. En dépassant la simple réflexion, autour d'un jeune homme plein de talent, nous avons décliné un mode d'action en soixante-trois préconisations pour la cité rurale. Elles ont vocation à ouvrir le champ des possibles. Je les tiens à votre disposition. Notre cité rurale, plutôt qu'une réponse définitive, vous propose un mode de réponse, en accord avec l'invite de Gérard Larcher : « La nation française constitue un héritage à partager, qu'il nous appartient de faire vivre et de transmettre. La cité rurale est de ces espaces qui engagent à ce partage. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons miser sur cette touche française qu'on nous envie, en prenant la ruralité comme un atout, une potentialité, et en y investissant, plutôt que d'y acheter temporairement une paix sociétale. le contraire serait renoncer à rester nous-mêmes et à notre ressource du troisième millénaire

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cette chambre haute qui représente au Parlement les territoires, le thème de ce débat sonne à la fois comme une espérance, une nécessité et une ambition politique. Disons-le sans ambages : la Nation se délitera, le pays se balkanisera, si nous continuons tous à tout miser sur les métropoles de notre pays pour répondre aux attentes de nos concitoyens vivant en zone rurale. Étant entendu qu'il nous faut aussi des métropoles dynamiques à taille européenne pour être présents dans la compétition internationale. Quelle place entendons-nous donner aux ruralités françaises pour la création de richesses économiques, sociales, environnementales et culturelles pour un développement durable dont le bien-être de chacun et l'intérêt général national doivent être les motifs premiers ? Il y a deux semaines, dans le cadre d'une procédure un peu surprenante,

sur le fond, ce texte technique a davantage traité du « comment » que du « quoi » ou du « pourquoi ». Nous avons été nombreux dans cet hémicycle à regretter que le remarquable travail du commissaire général à l'égalité des territoires, M. Morvan, ne soit pas exploité ou ne constitue pas le point d'entrée d'un vaste débat national sur la place et le rôle des ruralités en France. Pour l'avoir appréciée en tant que responsable d'exécutifs locaux hier, de sénateur aujourd'hui, je tiens à souligner la qualité du travail mené par le pour la rénovation urbaine en matière de renouvellement urbain. Nous jugerons dans la longue durée les effets de ces politiques, mais je pense que les principes structurants retenus sont adaptés aux enjeux. Dans la ruralité comme ailleurs, c'est l'économie qui fait la vitalité, le dynamisme du territoire. Or, tout au long des décennies passées, la productivité agricole a fait son oeuvre. Si l'objectif d'autosuffisance alimentaire à coût abordable pour le consommateur a été atteint, c'est au prix d'un double sacrifice : celui du revenu pour les agriculteurs, celui de la démographie pour les territoires. Dans notre République, où l'attachement des Français à l'égalité et à la justice se manifeste en ce moment de manière préoccupante, le darwinisme territorial et social n'est pas une option. Le sentiment d'abandon est une réalité dans de nombreuses campagnes. Que disait le Président de la République en juillet dernier devant le Congrès de Versailles ? Il en appelait à « une réorganisation de l'État à travers plus de présence sur les territoires », ajoutant : « Surtout, il faut enrayer un mode d'action publique qui a toujours procédé aux économies en réduisant sa présence sur les territoires. » Il nous disait croire à « l'installation de nouveaux projets », à un « rééquilibrage des territoires, par l'installation d'activités économiques, accompagnées, aménagées avec l'ensemble des élus locaux par le Gouvernement » et « un accompagnement des services de l'État dans le cadre de ce projet ». Sur le terrain, en réalité, nous constatons trop souvent l'inverse ... Tout, ou presque, reste à faire ! Dans quelque temps, nous examinerons le projet de loi sur les mobilités. Il faut que des réponses concrètes soient apportées aux Français des territoires ruraux qui sont et resteront captifs de la voiture pour vivre au quotidien. Je mesure tous les jours, au contact des entreprises installées dans le Gers ou qui voudraient s'y installer, les voies rapides et le rail restent des infrastructures majeures pour le développement économique et social. En particulier, il faut que l'État termine le plus vite possible les routes nationales, par lesquelles l'influence métropolitaine vitalise les territoires ruraux. Dès lors, monsieur le ministre, quelle est votre conception de la justice spatiale, un concept de plus en plus employé ? Quelle est votre définition de la cohésion des territoires, et sur quels critères la fondez-vous ? Comment, concrètement, doit se manifester la solidarité réciproque entre des territoires aux dynamiques très dissemblables, par exemple entre les métropoles et leurs zones rurales d'influence directe ou plus lointaine ? Quel rôle l'État doit-il jouer, dans le respect des principes de la décentralisation ? Souscrivez-vous à tout ou partie des propositions du rapport Morvan ? Bref, quels sont vos objectifs quantifiés pour gagner en cohésion territoriale ? Quelle est votre stratégie pour y parvenir, et suivant quel calendrier ? Quel processus au fil de l'eau prévoyez-vous pour évaluer l'efficacité de cette politique de cohésion des territoires ? Avec quelle implication- c'est une question importante -des élus et des citoyens ? Les élus locaux, tout particulièrement ceux des campagnes, désespèrent de pouvoir mener une action publique efficace et reconnue par leurs administrés. Ils ont besoin de respect, de visibilité, de stabilité, de moyens financiers propres et d'accompagnements divers, celui de l'État n'étant pas le moindre. Monsieur le ministre, pour que la ruralité soit une chance pour la France,

à l'heure où se tient le congrès de maires, permettez-moi de saluer ceux qui, par leur engagement et leur volonté de développer nos territoires, sont la preuve que la ruralité est une chance pour la France. Excusez-moi d'être un peu chauvine, mais je profite de cette occasion pour saluer les élus haut-pyrénéens présents en tribune ... C'est pour eux, qui font vivre C'est pour eux, qui font vivre nos territoires et leur offrent un cadre de vie unique, que mon groupe a fait le choix de ce débat, dont je me félicite. D'après un récent rapport de l'IFOP pour l'association Familles rurales, la vie à la campagne serait le mode de vie idéal pour 81 % des Français. Mieux, dans les territoires ruraux, nous connaissons une forte croissance de l'emploi, notamment des cadres. Ces chiffres démontrent clairement que la ruralité attire encore et se développe. Elle est le terreau fertile de valeurs ancrées dans notre identité, de traditions qui ont forgé notre image et dont les savoir-faire font la renommée internationale de notre pays. On connaît certes la France pour la tour Eiffel et ses musées, mais on l'aime aussi pour sa gastronomie, son patrimoine historique reconnu et admiré, pour les paysages variés et riches de ses 36 000 communes. Telle est la France : forte de ses villes, incomparable grâce à ses campagnes. Dès lors, reconnaître que la ruralité est une chance pour la France et traduire cela par des politiques de cohésion territoriale et de développement de tous les territoires, c'est redonner à notre pays les moyens de cette ambition. Voilà trop longtemps que les choix politiques font la part belle aux métropoles, privilégiant la concentration des pouvoirs décisionnaires et la raréfaction des services publics. Dans mon département, nous avons dû nous battre pour nos écoles, pour nos médecins, pour nos trésoreries et pour notre industrie. matière, les collectivités territoriales ont bien souvent pris le relais d'un État défaillant ou absent. À cela s'est ajoutée la loi NOTRe, qui a bouleversé les territoires. Fondée sur la politique du nombre, avec des critères démographiques contraignants, spécialement dans la ruralité, elle a modifié l'organisation des collectivités territoriales et concentré, encore et encore, les compétences. Alors que la commune reste dans nos territoires ruraux le dernier service public accessible aux citoyens, les intercommunalités mises en place à marche forcée par la loi NOTRe peinent toujours à s'organiser. Nous devons dès aujourd'hui entendre l'appel des maires, convaincus de la nécessité du maintien de ce lien entre nos concitoyens et nos institutions républicaines. Pour éviter un engrenage préjudiciable à la cohésion sociale, il nous faut continuer de faire de nos espaces ruraux des lieux de vie et de travail, par un aménagement du territoire renforçant leur attractivité. nous devons accompagner la forte croissance du télétravail pour attirer en ruralité les acteurs de l'économie numérique, sans exclure l'opportunité de renforcer le développement industriel. dans nos territoires les services publics de proximité, les commerces, les loisirs, une offre de santé adaptée et une offre culturelle et sportive riche. La cohésion territoriale, ce n'est pas, d'une part, des territoires qui concentreraient tout, de l'autre, des territoires vidés de tout service. Les Français doivent avoir le choix, et c'est à la République de le leur offrir : telle est l'idée que nous nous faisons de la France, indivisible et riche de ses diversités !

C'est comme si l'on se demandait si la médecine est une chance pour notre société, ou si la justice est une chance en démocratie- et demain, pourquoi pas, si c'est une chance que le soleil brille

ce sont ses racines et toutes les valeurs qui s'y rattachent ; elle est le creuset où s'est forgée notre identité, construite patiemment au fil des siècles. donc, la ruralité est une chance, mais elle fait intrinsèquement partie de notre territoire, et bien sûr de son développement. Depuis la nuit des temps, la ruralité existe dans tous les pays du monde, et je ne pense pas que cela va s'arrêter. nombre d'espaces autrefois en déshérence ont regagné de la population, qu'il s'agisse de jeunes couples, de retraités, d'agriculteurs, d'entrepreneurs ou de travailleurs indépendants pratiquant le télétravail, tous à la recherche d'une meilleure qualité de vie. de nouvelles perspectives et de nouveaux talents apportent un nouveau souffle et redonnent un destin à nos petites communes. Par ailleurs, ce sont les citadins eux-mêmes, à la recherche de leurs racines ancestrales, qui soignent le mieux l'habitat rural. l'habitat rural. Celui-ci devient une valeur refuge, une protection : face à toutes les tragédies que l'on peut lire dans la presse ou voir à la télévision, sur internet ou autrement encore, chacun recherche ses racines, et c'est pour cela que, dès qu'ils ont quelques jours, les gens des villes partent se réfugier, se détendre et se ressourcer à la campagne.

Il me semble pourtant que chacun apporte quelque chose à l'autre : les petits apportent beaucoup aux grands, car ce ne sont pas les richesses ou le paraître qui comptent, mais avant tout, en tout cas pour moi, la taille de notre coeur. Les gens de la périphérie n'hésitent pas à prendre des risques et, même dans les moments difficiles, ne baissent pas la tête ; ils ne renoncent pas, car ils veulent que la prochaine génération et les suivantes vivent dans un monde bien meilleur. Vu qu'ils ont moins de moyens et de sollicitations extérieures, ils font preuve d'une ingéniosité et d'une créativité plus grandes, innovant pour atteindre à l'excellence. D'ailleurs, tout le monde sait fort bien que de nombreuses personnalités illustres sont issues du monde rural. La ruralité est une niche de pépites, tout comme l'outre-mer : c'est une richesse, une ouverture sur le monde et d'autres horizons. De nombreuses études montrent aujourd'hui à quel point les communes rurales, pourtant loin d'être majoritaires en population, pèsent dans la dynamique économique du territoire national. Preuve que rien n'est perdu, si l'on utilise les bons leviers Ce dont ont besoin tous les acteurs ruraux, c'est d'un formidable coup de pouce à l'activité : allégement des charges et de la fiscalité, simplification drastique des normes et règlements qui étouffent les PME. Comme les maires de nos petites communes, arrêtons de vouloir laver plus blanc que blanc. Relançons l'apprentissage et la formation professionnelle. Le voilà, l'oxygène de nos campagnes Les territoires ruraux ne demandent pas l'aumône. Non, l'État se doit d'écouter, d'entendre et d'agir, d'agir vite, car ces territoires sont remplis d'atouts à développer. Arrêtons donc de traiter les territoires ruraux comme un repaire de rats des champs devant muter en rats des villes pour survivre, et envisageons réellement ces territoires non comme une chance, mais comme un levier indispensable pour notre économie et comme une continuité avec les villes.

vais m'y efforcer ... Monsieur le ministre, mes chers collègues, la ruralité est un véritable atout pour la France. En effet, nos campagnes font partie intégrante de notre identité française : elles représentent près de 80 % du territoire, et un habitant sur cinq y réside aujourd'hui. L'exceptionnelle diversité des paysages français et le patrimoine culturel qu'ils représentent font de ces territoires une source incontestable de qualité de vie. D'après un récent sondage, pour plus de 80 % des Français, vivre à la campagne représente la vie idéale, qu'ils y travaillent ou non. Comment parler de la ruralité sans évoquer nos agriculteurs ? Soucieux de leur environnement, conscients de leur potentiel économique, ils façonnent nos paysages et font rayonner les produits français à travers le monde. Depuis peu, les flux migratoires observés en France entre milieu rural et milieu urbain s'inversent progressivement les derniers recensements font apparaître l'inversion de la migration des départements ruraux vers les départements urbains. Même s'ils ne concernent qu'une partie de la population, flux sont suffisants pour provoquer l'accroissement de nombreuses communes rurales des départements français. Bien entendu, ces mouvements sont très diversifiés et touchent de façon inégale les diverses parties du territoire. Nous observons depuis quelques décennies un regain d'appétence pour nos territoires ruraux. La qualité de vie, le calme et la nature apparaissent comme les principaux attributs de la ruralité qui conduisent des Français à s'installer à la campagne. Mes chers collègues, nous devons mettre en oeuvre tous les moyens pour que les opportunités économiques deviennent un argument supplémentaire. Bien entendu, la santé, les services de proximité et la mobilité sont des conditions prioritaires pour l'attractivité et le développement des zones rurales.

Dès le début de son mandat, le Président de la République a fixé le cap : développement du haut débit en 2020, puis du très haut débit en 2022. Il est primordial d'atteindre ces objectifs. En effet, c'est en résorbant la fracture numérique entre milieu urbain et milieu rural que nous redynamiserons nos campagnes. Quand on n'a pas accès au numérique, on n'a pas accès aux opportunités », comme l'a déclaré le secrétaire d'État chargé du numérique en juin dernier. Une multitude d'acteurs économiques du tertiaire, cantonnés aujourd'hui aux centres-villes et aux périphéries urbaines, constituent un formidable potentiel pour l'implantation de nouvelles activités économiques en zone rurale, notamment à travers de nouveaux phénomènes professionnels comme la numérisation des relations de travail et l'auto-entrepreneuriat. Profitons de la tendance migratoire que je viens de décrire pour amplifier cet exode urbain, encore marginal, qui permettrait une meilleure qualité de vie pour les néo-ruraux, un désengorgement significatif de nos villes et des zones sous tension et une redynamisation redynamisation de la vie sociale de nos territoires ruraux. Cet exode rural ne sera possible que si les objectifs de couverture numérique et de fin des zones blanches sont atteints, et que le développement du télétravail en milieu rural est soutenu.

Comment le Gouvernement compte-t-il tenir ses promesses en termes de couverture numérique pour résorber la fracture en la matière ? Parallèlement au déploiement de la couverture numérique, prévoit-il des mesures d'accompagnement,

Si plus de 20 millions de Français vivent dans ces territoires, soit un tiers de la population française, si le nombre d'habitants dans les territoires ruraux augmente plus vite que dans les centres urbains, si le solde migratoire y reste encore positif, c'est bien parce que les Français aiment ces territoires, veulent y vivre, y travailler, y élever leurs enfants, car ils trouvent dans cette France rurale une qualité de vie incomparable, et ce malgré les promesses que les métropoles peuvent représenter. Au fond, ces quelques chiffres illustrent tout le paradoxe de la ruralité. Nos concitoyens plébiscitent la campagne, les ruralités, ils veulent majoritairement y vivre, et, dans le même temps, la représentation des ruralités dans le débat public reste connotée négativement c'est la France périphérique, celle de territoires qui se sentent oubliés et qui seraient nécessairement les victimes de la globalisation et de la métropolisation. Le Gouvernement, comme chacun ici, veut sortir de cette vision manichéenne, parfois défaitiste, lorsqu'il est question de ces territoires. Ce discours, nous devons le refuser collectivement, car il nourrit une image qui n'est en rien fidèle aux richesses des territoires ruraux, au dynamisme et au potentiel de leurs habitants, à leur capacité d'innovation et aux valeurs qui les animent. Mais en même temps nous devons regarder en face les difficultés qui existent et persistent. Nous ne devons pas éluder le fait que certains territoires ont perdu ces dernières années parfois plus d'un quart de leurs emplois et finalement une part significative de leur population, et que, lorsque la démographie chute, ce sont les commerces et dans le même temps les services publics qui disparaissent. Oui, il existe, dans certains territoires ruraux un vrai sentiment d'abandon, comme l'a souligné Franck Montaugé. Oui, il existe une idée selon laquelle la République aurait décidé de regarder ailleurs, privilégiant les grandes villes. C'est bien cela, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement ne compte plus accepter. C'est pourquoi depuis dix-huit mois le Gouvernement s'est pleinement mobilisé en faveur des territoires ruraux en faisant appel aux moyens propres de l'État. Cette mobilisation n'est pas une simple incantation. C'est un objectif qui se traduit en actes. J'en donnerai quelques exemples. Sur le plan financier d'abord, nous maintenons au plus haut niveau les dotations de soutien à l'investissement en faveur des territoires ruraux. La DETR a ainsi augmenté de 400 millions d'euros par rapport à 2014 pour atteindre plus de 1 milliard d'euros en 2019. De même pour la DSIL, qui reste au niveau des années précédentes alors qu'elle était au départ

L'accompagnement financier, s'il est indispensable, ne suffit pas. C'est pourquoi le Gouvernement est allé plus loin. En effet, faire plus pour ceux qui ont moins, cela signifie, s'agissant des territoires ruraux les plus vulnérables- ceux qui cumulent les plus fortes difficultés économiques, sociales, démographiques -, qu'il faut prévoir un accompagnement spécifique actionnant tous les leviers

même de petite taille, a toujours un effet d'entraînement sur les territoires avoisinants. Aussi, quand le Gouvernement engage le programme Action coeur de ville- je salue Jacques Mézard, qui en est à l'initiative -en mobilisant 5 milliards d'euros sur cinq ans au profit de deux pour réhabiliter des logements, réimplanter des commerces et rénover les espaces publics, il agit aussi pour les territoires ruraux qui vivent en symbiose avec la ville voisine. Soutenir les territoires ruraux, c'est également garantir la présence des services au public dans ces territoires. C'est tout le sens des 1 300 maisons de service au public qui ont été lancées par le précédent gouvernement et que nous continuons de déployer. Pour ce qui concerne la réforme de l'État territorial, le Premier ministre détaillera prochainement son contenu. Mais les principes qui guident cette réforme sont ceux de l'État de proximité, car l'État ne peut se vivre au seul niveau régional et doit s'incarner au plus près des habitants.

; création d'une prime pour encourager la réalisation de stages de médecine dans les zones qui rencontrent des problèmes de démographie ; déploiement de 400 médecins salariés dans les déserts médicaux ; accélération des maisons de santé pluridisciplinaires ; renforcement des hôpitaux de proximité ; remboursement pour tous de la télémédecine grâce à un accord avec l'assurance maladie ; déploiement, d'ici à 2022, de 1 000 communautés professionnelles territoriales de santé. Le service public, c'est aussi l'éducation nationale, comme l'a rappelé Cécile Cukierman. C'est pourquoi 400 postes supplémentaires seront créés en deux ans dans les quarante-cinq départements les moins denses, qui viendront s'additionner aux mesures déjà déployées et qui ont permis d'accroître le taux d'encadrement des élèves sur l'ensemble du territoire, notamment dans les départements les plus ruraux.

Le Gouvernement n'accepte pas que des pans entiers de nos territoires soient coupés du monde, dans des « zones blanches », qui interdisent l'accès à une part significative de l'information disponible et qui freinent le développement des entreprises ... Monsieur le ministre, il vous reste trente secondes.

les besoins alimentaires qui restent importants, en particulier dans un contexte de dérèglement climatique ; les besoins énergétiques nouveaux rappelés par certains d'entre vous ; les besoins fonciers pour peu qu'ils soient moins subis par les territoires et davantage voulus. Pour ce faire, nous devons conjurer plusieurs risques. Celui du et de la culture d'une nostalgie,

en déposant cette proposition de loi organique, il y a quelques semaines, je n'imaginais pas un instant qu'elle susciterait autant de réactions, voire autant de passions. J'entends bien la conviction profonde qui habite nombre d'entre vous et qui consiste à penser que, pour prétendre devenir sénateur, il conviendrait au préalable d'avoir exercé un mandat d'élu local. Quelle horreur ! Notre Constitution qualifie en effet notre assemblée de « chambre des territoires », et tout au long de son histoire celle-ci s'est toujours posée en défenseur des collectivités locales. Sachez, mes chers collègues, que je respecte cette conviction et que je ne vise pas à la contester par ce texte. Il ne s'agit ici que d'une proposition de loi visant à assurer la cohérence de notre droit interne au regard du droit désormais commun dans notre pays à toutes toutes les élections. Dans toutes les démocraties consolidées comme la nôtre, l'heure est en effet à l'universalité de plus en plus étendue de l'éligibilité concernant les fonctions sujettes à mandat électoral. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, qu'en 2011 nous avons abaissé à dix-huit ans l'âge d'éligibilité à l'élection présidentielle, de même que celui de nos députés. Cependant, nous nous doutons bien, au regard des attentes de nos concitoyens et de leurs pratiques de vote, que l'élection d'un Président de la République de moins de vingt-cinq ans a très peu de chance de se produire un jour. Aussi, dans ce débat sur l'âge d'éligibilité, la logique et la raison doivent absolument l'emporter sur la conviction et sur l'émotion. Il faut donc bien veiller à ne pas confondre accès à un droit et effet produit par ce droit dans les faits. Être éligible et être élu représentent deux choses bien distinctes, même si, naturellement, pour être élu, il faut être éligible. C'est le droit qui définit l'éligibilité, mais ce sont les électeurs qui choisissent les élus. Mes chers collègues, c'est précisément votre esprit de logique et de cohérence- propre à votre fonction de législateur -que je sollicite en tentant de vous démontrer que le seuil de vingt-quatre ans, aujourd'hui en vigueur, est à la fois inéquitable, inéquitable, incohérent et inutile. Inéquitable, tout d'abord, car la règle actuellement en vigueur exclut plus de 4 millions de jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, dont certains sont des élus locaux ou des grands électeurs lors des élections sénatoriales. Dans mon bon département des Hauts-de-Seine, ils n'étaient pas moins de trente-huit dans cette situation lors du renouvellement sénatorial de l'an passé, grands électeurs, obligés de voter sous peine d'amende en cas de manquement, mais interdits de figurer sur une liste sénatoriale, même en position de suppléant. L'existence d'un âge minimal d'éligibilité supérieur à l'âge de la majorité est injuste, voire dangereuse, car elle ouvre la voie par parallélisme à une possible fixation d'un âge maximal d'éligibilité.

au regard des règles générales d'éligibilité en vigueur lors de toutes les autres élections ouvrant droit à mandat public dans notre pays, et même pour la plupart des grandes fonctions de l'État : ministre, membre du Conseil constitutionnel ou encore, et dans un autre registre, membre du Conseil économique, social et environnemental.

À ce stade de notre réflexion, il serait intéressant, je crois, de nous pencher sur l'exemple de la Belgique et sur les conditions d'éligibilité en vigueur dans ce pays en matière d'élections sénatoriales. Alors qu'en 1993 le Parlement belge avait déjà abaissé de quarante à vingt et un ans l'âge d'éligibilité au Sénat, une chambre désignée au suffrage universel indirect par les représentants des territoires qui composent la fédération, nos collègues belges ont en 2014 procédé à un nouvel abaissement de ce seuil à les raisons invoquées pour justifier cette nouvelle réforme ? Dans leurs attendus, nos collègues belges ont procédé à cet abaissement, car ils jugeaient « raisonnable et objectivement justifié de prendre cette mesure dès lors que l'âge de dix-huit ans est demandé pour toute élection en Belgique ». Ils ont également invoqué « une rupture du principe d'égalité en cas de non-alignement de l'âge d'éligibilité des parlementaires sur celui concernant les autres mandats électifs ». Monsieur le président de la commission des lois, vérité outre-Quiévrain, erreur en deçà ? Enfin, concernant toujours les principes d'égalité et de cohérence de notre droit électoral, je rappelle que, conjointement avec l'Assemblée nationale, la Haute Assemblée constitue le parlement de la France. France. Dans ce cadre, nous pouvons être appelés à nous réunir en Congrès pour prendre des décisions majeures pour notre pays. Aussi, si rien n'oblige à avoir le même mode de scrutin et le même corps électoral dans les deux chambres, il est en revanche très discutable, en termes de droit d'accès à l'élection, de ne pas disposer des mêmes règles d'éligibilité.

Nous disposons heureusement du même champ de compétences que l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas pour tous les sénats dans le monde. Notre spécificité de « chambre des territoires » repose, d'un point de vue juridique et législatif, exclusivement sur la nature du corps électoral appelé à nous élire. Le choix d'un sénateur obéit donc à des critères fixés par les grands électeurs, souverains en la matière. Adjoindre à ce processus un critère d'âge spécifique, c'est exprimer une forme de défiance à l'endroit du jugement de nos grands électeurs. Bref, cette condition d'âge, ajoutée à la nature spécifique du corps électoral du Sénat et de ses modalités de scrutin, fait un peu, mes chers collègues, passez-moi l'expression, « ceinture et bretelles » ! À ceux qui disent qu'un abaissement du seuil d'âge d'éligibilité reviendrait à dénaturer notre Sénat, je veux leur dire sans emphase : « n'ayez pas peur ! » La meilleure des preuves, c'est celle qui relève des faits observés. L'abaissement en 2011 de l'âge d'éligibilité de trente à vingt-quatre ans n'a pas provoqué de bouleversement sociologique et démographique au sein du Sénat. Lors des trois renouvellements

argument souvent avancé pour ne pas abaisser davantage l'âge d'éligibilité au Sénat : nombre d'autres hautes chambres en Europe, et ailleurs, fixent elles aussi un âge d'éligibilité de leurs représentants supérieur à l'âge légal de la majorité. C'est vrai, mais elles sont de moins en moins nombreuses. De plus, ce seuil, quand il existe, répond souvent à des considérations très particulières liées aux spécificités des modes de scrutin ou de désignation desdites chambres.

! Si l'on se penche uniquement sur le cas des treize États disposant d'un Parlement bicaméral, six d'entre eux, et non des moindres-l'Allemagne, l'Espagne -disposent d'un seuil d'éligibilité à dix-huit ans pour leur sénat et deux autres établissent celui-ci à vingt et un ans. Sur les cinq pays restants, dont la France, quatre- l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque -disposent d'un sénat élu au suffrage universel direct, le plus souvent le même jour que la tenue des élections législatives. dans ces pays, la fixation d'un seuil d'éligibilité plus élevé est le seul critère permettant de différencier la composition de la Haute Assemblée de celle de la chambre basse. Alors, oui, la France fait bien figure d'exception dans le concert des parlements nationaux au sein de l'Union européenne, puisque c'est le seul pays bicaméral où un Sénat élu au suffrage universel indirect, suivant un mode de scrutin très différent de celui de l'Assemblée nationale et à des dates bien distinctes de celle-ci, s'autorise, de surcroît, à fixer un seuil d'éligibilité de six ans supérieur à celui de la chambre basse. Vous le voyez, mes chers collègues, tout dans cette proposition de loi organique n'est qu'affaire d'équité, de cohérence et aussi de reconnaissance de la légitimité de chacun à espérer concourir à la représentation de la Nation. À l'heure où la représentation nationale et le Sénat en particulier sont trop injustement vilipendés dans l'opinion, l'abaissement de l'âge

Ce seuil de vingt-quatre ans a été défini pour donner l'opportunité aux sénateurs, représentants des collectivités territoriales au sens de l'article 24 de la Constitution, d'exercer un mandat local avant d'entrer au Palais du Luxembourg. La proposition de loi organique n° 744 relative à l'élection des sénateurs, présentée par notre collègue André Gattolin, a pour objet de réduire l'âge d'éligibilité des sénateurs de vingt-quatre à dix-huit ans pour plusieurs raisons. il s'agit de faire concorder l'âge d'éligibilité avec la citoyenneté. Deuxièmement, il s'agit de simplifier les règles pour que l'âge d'éligibilité soit à dix-huit ans pour toutes les élections. Troisièmement, parce qu'un mandat d'élu local n'est pas indispensable pour faire un bon sénateur.

Dans le rapport, nous avons souhaité rappeler le rôle du Sénat, ses spécificités et les objectifs à atteindre. Le Sénat est une haute assemblée qui a trois missions : voter la loi, contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques. Mais le Sénat assure aussi la représentation des collectivités territoriales et des Français établis hors de France. Conformément à la Constitution, l'équilibre de la VRépublique repose sur un bicamérisme différencié, mais équilibré. Il est primordial d'avoir et de conserver deux chambres différentes et complémentaires. Pour ce faire, deux modes de scrutin différents ont été instaurés pour le Sénat et l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, l'âge d'éligibilité est fixé à vingt-quatre ans et diffère de celui des députés. Le scrutin est majoritaire, dans les circonscriptions comportant jusqu'à deux sénateurs, ou de liste dans les autres. Enfin, le mandat dure six ans avec un renouvellement partiel tous les trois ans. Comme l'a récemment déclaré notre collègue Philippe Bas et comme le démontre l'actualité récente, « le Sénat constitue ainsi un pouvoir non aligné, libre et indépendant ». En effet, « le mode d'élection des sénateurs, leur enracinement dans nos collectivités sont pour la démocratie une garantie de liberté et de pragmatisme

À l'époque, déjà, la chambre haute devait concilier l'évolution du régime tout en maintenant la paix sociale. L'âge était perçu comme un facteur de modération et de valorisation des expériences locales. Le général de Gaulle a d'ailleurs déclaré lors du discours de Bayeux que « le premier mouvement- de l'Assemblée nationale -ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération ».

En outre, nous sommes les représentants des collectivités territoriales. Comment est-il possible de représenter sans connaître le fonctionnement de ces collectivités ? Certes, certains sénateurs n'ont pas exercé de mandats locaux, mais ils sont rares. Ces mêmes sénateurs peuvent exercer leur mandat en excellant dans des sujets autres de sociétés. Mais si tous les sénateurs sont dans le même cas, alors les collectivités territoriales perdront leur confiance dans le Sénat, considérant que ce dernier est loin de leurs préoccupations comme la revitalisation de l'échelon communal, la GEMAPI ou les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. Il est donc indispensable de maintenir l'âge d'éligibilité de vingt-quatre ans pour s'assurer que les sénateurs seront choisis par les grands électeurs, parce qu'ils ont accompli un mandat local et parce qu'ils ont l'expérience suffisante et nécessaire pour garder le statut de représentant des collectivités. Les débats de 2011 démontrent d'ailleurs que l'âge de vingt-quatre ans a été défini en additionnant l'âge de la citoyenneté et la durée d'un mandat local complet. Faut-il diminuer l'âge d'éligibilité à dix-huit ans pour rajeunir l'âge moyen des sénateurs ?

Les âges moyens entre les deux assemblées étaient assez proches. Je parle à l'imparfait, car il y a eu les dernières élections législatives ! L'écart s'est creusé, puisque la moyenne d'âge des députés est passée à quarante-neuf ans et celle des sénateurs est restée à soixante

Notre collègue André Gattolin reconnaît d'ailleurs qu'il est peu vraisemblable que des sénateurs âgés de dix-huit à vingt-quatre ans soient élus, sauf sur des scrutins de liste. Leur nombre étant limité, cela n'influencera pas la moyenne d'âge. On s'est alors interrogé sur le but recherché au travers du rajeunissement de la Haute Assemblée. Serait-ce utile pour aborder des sujets concernant la jeunesse dont on ne traiterait pas aujourd'hui ? Les décisions sont-elles adaptées à toutes les générations ? Pour répondre à ces questions, nous avons auditionné nos plus jeunes députés sur leur fonction et la représentativité de leur génération. Ils nous ont démontré qu'ils n'étaient nullement spécialisés dans ces sujets et que leurs opinions ne différaient pas, ou peu, de celles de leurs collègues sur l'ensemble des textes. La jeunesse était un sujet abordé, suivi et pris en considération par des élus qui étaient en contact avec ces générations et qui avaient de l'intérêt pour ces À titre d'exemple, le Sénat est intervenu sur l'obligation de transparence des algorithmes utilisés dans Parcoursup pour classer les étudiants ... Enfin, sommes-nous différents des autres pays ? Non ! Seules l'Allemagne et l'Espagne ont fait le choix d'avoir des âges identiques dans les deux chambres. Mais il est difficile de se comparer à l'Allemagne, puisque les membres du Bundesrat sont désignés par le gouvernement de leur Il est clair que tous les autres pays ont fait le choix de maintenir la différence des âges, notamment les États-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Peut-on aborder cette proposition de loi organique sans prendre en considération les projets du Gouvernement concernant la réforme de nos institutions ? Ces projets pourraient d'ailleurs remettre en question les spécificités du Sénat, en multipliant par quatre le nombre de départements ne comptant qu'un seul sénateur en supprimant, pour les prochaines élections sénatoriales, le principe du renouvellement partiel au bénéfice d'un renouvellement intégral du Sénat en 2021. Comme l'a déclaré notre collègue Jérôme Bignon lorsqu'il était député en 2003 : « La différence d'âge [entre les deux chambres] est une richesse. N'uniformisons pas les mandats, les modes d'élection et les périodes de renouvellement, car nous risquerions de sombrer dans un bicamérisme affadi. » En conclusion, j'émets un avis défavorable sur la proposition de loi organique qui tend à réduire l'âge d'éligibilité des sénateurs de vingt-quatre En effet, il me semble préférable de maintenir une différence d'âge entre les deux assemblées, avec un mode d'élection différent, pour que la chambre haute fasse toujours preuve de sagesse pour relire, instruire, négocier et débattre des propositions de lois votées en première lecture. ailleurs, le Sénat est le représentant des collectivités. Les sénateurs perdront toute crédibilité s'ils n'ont pas exercé de mandat dans ces collectivités et s'ils n'ont pas l'expérience nécessaire. Il peut y avoir une proportion de sénateurs sans mandat qui exercent brillamment, mais celle-ci doit être limitée.

Plus globalement, nous ne pouvons pas faire abstraction du débat en cours sur la réforme des institutions. L'âge est un élément essentiel, qui doit être abordé avec l'ensemble

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur Gattolin, mesdames, messieurs les sénateurs, la présente proposition de loi organique vise à réduire à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au mandat de sénateur.

Je concentrerai mon propos sur trois éléments qui fondent la position du Gouvernement sur cette proposition de loi organique. Premièrement, aucun obstacle juridique et aucun principe constitutionnel ne s'opposent à l'abaissement à dix-huit ans du seuil d'éligibilité au mandat sénatorial. Autrement dit, il s'agit là d'une question d'opportunité. L'engagement présidentiel en la matière est celui du renouvellement de la classe politique et d'une plus grande place faite à la jeunesse. C'est pour cette raison que le Gouvernement ne peut être que favorable à cette proposition de loi. Comme vous l'avez rappelé, monsieur Segouin, dans votre rapport fait au nom de la commission des lois, les régimes d'éligibilité ont été progressivement harmonisés au fil des années, de sorte que si l'on excepte les cas particuliers du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'élection sénatoriale, tous les scrutins français sont désormais accessibles dès l'âge de Le seuil d'éligibilité au mandat de conseiller municipal a été abaissé à dix-huit ans dès 1982. Celui pour les élections départementales et régionales l'a été en 2000. Enfin, la loi organique du 14 avril 2011 a abaissé à dix-huit ans le seuil d'éligibilité aux mandats présidentiel, de député et de député européen. L'abaissement à dix-huit ans de l'âge d'éligibilité au Sénat va donc dans le sens de l'harmonisation et de la simplification du droit. Cette évolution permettra d'aligner, pour tous les tous les scrutins, l'âge d'éligibilité avec l'âge d'exercice du droit de vote, un des premiers droits fondamentaux de chaque citoyen, qui est aussi un devoir, celui de participer à la vie de la cité. Actuellement, nous demandons à des citoyens- grands électeurs en l'occurrence -de participer à la désignation de leurs représentants, mais une partie d'entre eux n'auraient pas le droit de candidater, étant trop jeunes. Je crois que vous avez raison, monsieur le sénateur Gattolin, en soulignant que cette situation, qui est certes un héritage de l'histoire, pourrait être amenée à évoluer. Deuxièmement, le Sénat assure la représentation des collectivités locales. C'est effectivement l'une des missions que lui confie la Constitution, et elle est essentielle. Nous en avons tous conscience, car dans notre République, dont l'organisation est décentralisée, les collectivités territoriales ont leur mot à dire. Mais je ne suis pas convaincu qu'il soit absolument nécessaire d'avoir exercé un ou plusieurs mandats pour représenter avec fidélité les collectivités. Ce qui fait l'ancrage local des sénateurs, c'est aussi le mode de scrutin, autrement dit l'élection au suffrage universel indirect et la composition du collège électoral et la circonscription d'élection.

n'aura pas pour effet de transformer le Sénat en « clone » de l'Assemblée nationale, comme j'ai pu le lire et l'entendre. Si ! Le Gouvernement est attaché au bicaméralisme. Les réformes institutionnelles que nous entendons mener ne le remettent pas en cause. Par ailleurs, sur ce point, je pense que nous sommes tous d'accord ici pour convenir que cette évolution ne va pas conduire à un bouleversement sociodémographique du Sénat. Les précédents abaissements du seuil d'éligibilité n'ont pas été sans effet, mais cet effet est resté limité, il faut le reconnaître. La moyenne d'âge des sénateurs est relativement stable dans le temps, et je doute que l'élection d'un ou deux sénateurs de moins de vingt-quatre ans modifie « l'ADN » du Sénat. Dès lors, pourquoi refuser l'entrée à quelques personnalités qui ont probablement beaucoup à apporter aux travaux du Sénat si le collège électoral, composé de grands électeurs, responsables, estime qu'elles méritent ce mandat ? Cela m'amène à mon troisième et dernier point : le besoin de renouvellement. Le gouvernement auquel j'appartiens est attaché à ce principe, non pas par dogmatisme, mais parce qu'il est essentiel à notre démocratie et à la confiance de nos concitoyens dans le système politique. C'est pour cela que nous portons et que nous défendons l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, dispositions intégrées aux projets de loi organique et ordinaire que vous aurez à examiner prochainement. C'est aussi pour cela que nous sommes favorables à toutes les initiatives parlementaires visant à favoriser l'engagement des jeunes et leur accès aux responsabilités politiques. La proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui s'inscrit, bien sûr, dans cette logique. Si, comme je l'ai rappelé, ses effets seront limités, ils ne seront pas nuls. Jusqu'en 2003, l'âge minimum pour devenir sénateur était fixé à trente-cinq ans. Quatre sénateurs représentant diverses sensibilités ne seraient pas parmi vous aujourd'hui si ces dispositions étaient encore applicables. Je suis enfin assez réservé quant à l'affirmation selon laquelle l'âge est synonyme de modération. Si le Gouvernement est tout à fait conscient des spécificités du Sénat sur ce point, il est beaucoup moins convaincu par l'idée selon laquelle cette hauteur de vue serait liée au maintien d'une barrière d'accès à vingt-quatre ans. Sénat tient surtout à son mode de renouvellement, par moitié tous les trois ans, ainsi qu'à la durée du mandat sénatorial, six ans, lequel n'est pas corrélé aux cycles présidentiel et législatif. Aucun de ces points fondamentaux n'est remis en cause par la présente proposition de loi Enfin, j'en viens à la raison principale qui a été évoquée par la commission des lois pour motiver son rejet du texte. J'entends l'argument selon lequel ce sujet devrait être traité de manière globale, lors de l'examen des projets de loi organique et ordinaire pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Les sujets peuvent à première vue apparaître liés. Néanmoins, les textes présentés par le Gouvernement répondent à un engagement présidentiel fort, exprimé lors de la campagne électorale de 2017. La question de l'âge d'éligibilité des sénateurs n'a pas été évoquée dans ce cadre et n'a donc pas été intégrée dans le projet de loi organique que le Gouvernement porte. Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir qu'une initiative parlementaire conduise à l'ouverture de ce débat. Il ne m'appartient pas ici de défendre dans le détail des projets de loi qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée. Le temps de l'examen de ces réformes institutionnelles viendra. Néanmoins, je crois pouvoir affirmer qu'aucun de ces textes, qu'il s'agisse du paquet institutionnel porté par le Gouvernement ou de la proposition de loi déposée par le sénateur Gattolin,

depuis 2011, l'âge d'éligibilité des candidats aux élections sénatoriales est fixé à vingt-quatre ans, alors que celui des candidats aux autres élections a été abaissé à Ce seuil de vingt-quatre ans a été défini pour donner l'opportunité aux sénateurs, représentants des collectivités territoriales au sens de l'article 24 de la Constitution, d'exercer un mandat local avant d'entrer au Palais du Luxembourg. La proposition de loi organique relative à l'élection des sénateurs que nous examinons a pour objet de réduire l'âge d'éligibilité des sénateurs de vingt-quatre à dix-huit ans. Ce texte appelle plusieurs remarques. En premier lieu, il est nécessaire d'avoir un minimum d'expérience pour pouvoir exercer le mandat de sénateur. C'est tautologique ! À cet égard, l'enracinement local est fondamental, car il nous permet d'être proches des réalités concrètes des collectivités territoriales dont nous sommes les représentants. L'expérience de la gestion locale nous donne un éclairage particulier et irremplaçable sur la réalité sociale qu'aborde l'action politique. Cette expérience locale est plus que nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner des problématiques aussi spécifiques que les zones de revitalisation rurale, les services publics de proximité ou la ou la revitalisation de l'échelon communal, qui a donné lieu à un excellent rapport que nous venons de publier. En deuxième lieu, l'abaissement de l'âge d'éligibilité pourrait entraîner une inégalité de représentation dans nos territoires. À titre d'exemple, le département de l'Aveyron comprend deux sénateurs élus au scrutin uninominal. Or un candidat de dix-huit ans n'aurait véritablement de chance d'être élu qu'au scrutin proportionnel, dans les départements les plus peuplés et non en zone rurale. En troisième lieu, cette proposition de loi organique ne peut pas être examinée indépendamment des projets, plus larges, de réforme institutionnelle. En effet, le Gouvernement a déposé en mai dernier trois projets de loi « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace ». Le premier texte relève du domaine constitutionnel, le deuxième du domaine organique et le dernier de la loi ordinaire. Or ces projets de loi comportent plusieurs dispositions qui pourraient remettre en cause les spécificités du Sénat, mais également l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. il apparaît logique que l'ensemble de ces sujets soient examinés conjointement, dans le cadre d'un débat plus large sur les réformes institutionnelles et l'avenir du bicamérisme.

notre collège André Gattolin, soutenue par notre groupe, est en tout point conforme à la sagesse sénatoriale, et fidèle à cette sagesse qui procure à notre assemblée sa légitimité institutionnelle. Mais peut-être sommes-nous dans l'erreur Il n'est pas impossible, en l'espèce, qu'elle contienne en creux quelques éléments contrevenant à une certaine idée du Sénat. Auquel cas, si des arguments de cette nature nous étaient avancés, croyez bien que nous les examinerions avec la sagesse qui nous aurait jusqu'ici fait défaut. Mais c'était sans compter sur la vigilance sans faille de notre honorable commission des lois, qui a su déconstruire de bout en bout la logique fallacieuse de notre raisonnement. Grâce à elle, la République l'a échappé belle : la proposition de loi organique a été rejetée et, avec elle, l'abaissement de l'âge d'éligibilité fortement compromis. Au motif qu'elle galvaudait les formes élémentaires du bicaméralisme, une fin de non-recevoir lui a été opposée, sans autre forme de procès, si ce n'est quelques arguments qui nous ont fait l'effet d'un attrape-mouche savamment élaboré. Mais peut-être qu'à la faveur d'un examen de conscience, notre cher rapporteur, de ligne de conduite et se ralliera aux tenants de cette disposition organique, fût-ce au prix d'une désaffiliation partisane. Après tout, comment pourrait-il en être autrement ? Comment autrement ? Comment une chambre parlementaire comme la nôtre, en proie à des procès en représentativité sans cesse plus sévères, pourrait-elle se réfugier dans une forme d'inertie ? Comment des sénateurs de bonne foi, sous le joug de calomnies imméritées, au gré desquelles les partisans d'un monocamérisme anémique gagnent du terrain, pourraient-ils refuser cette mesure de bon sens ? Mes chers collègues, cette appréciation négative portée sur l'action de notre institution ne doit pas faire taire notre apport substantiel à la machine parlementaire, dont notre honorable assemblée tire son sens et sa fonction. Nous devons d'instinct nous faire l'écho d'une institution à l'écoute des évolutions sociétales, comme l'a dit très justement mon ami André Gattolin. Admettons un instant que le législateur organique refuse cette proposition, dont l'évidence s'impose d'elle-même. Imaginez maintenant que cette assemblée, en vertu de je ne sais quel principe juridique, oppose à ses détracteurs les plus forcenés un esprit corporatiste de circonstance. Pis encore, que les commentaires médiatiques réceptionnent grossièrement le vote d'aujourd'hui comme une manoeuvre identitaire de mauvais aloi. Ce vote nous ferait-il l'effet d'un Sénat étranger à lui-même pour qui la sagesse ne serait qu'une chimère de plus ? Or, mes chers collègues, l'on ne s'y trompe pas, l'alignement sur le droit commun de l'âge d'éligibilité spécifique aux élections sénatoriales n'est guère autre chose qu'une mesure de sagesse. Sans être fidèle à un quelconque esprit démagogique,

l'âge d'éligibilité ? L'identité sénatoriale en réchapperait-elle ? Nous en sommes intimement convaincus. Cela étant dit, l'inverse est encore moins sûr. Je suis même tenté d'aller plus loin : votre conception de l'éligibilité nous semble, sous bien des rapports, contraire au principe d'égalité, tant et si bien qu'elle ne saurait prospérer en l'absence de justifications politiquement indiscutables. Ces justifications, parlons-en ! Lorsqu'elles ne sont pas desservies par une physionomie passablement ringarde, nous sommes bien en peine de les trouver. Voici quelques éléments de précision. D'abord, sur la douteuse nécessité d'acquérir, avant toute implication législative, une certaine expérience locale des mandats politiques, logique qui présida il y a peu à la détermination du seuil des je vais vous dire mon sentiment : la jeunesse n'est qu'un mot, mais c'est aussi le guet-apens par excellence. Ne tombons pas dans l'ornière des préjugés. Si nous le faisons, il n'est pas certain que la sagesse des vieilles troupes, que l'on peut constater sans réserve dans nos rangs, soit toujours le gage d'un travail parlementaire et législatif dûment mené tout juste y contribue-t-elle. En outre, André Gattolin l'a rappelé, l'âge d'éligibilité pour être Président de la République étant de dix-huit ans, faut-il en conclure qu'une sagesse plus prodigieuse encore est nécessaire pour souscrire aux conditions d'éligibilité de l'élection sénatoriale ? Un tel examen de capacité vise-t-il à se prémunir contre une jeunesse bien-pensante aux dents longues et aux idées courtes ? Plus sérieusement, l'argument ne tient pas à l'examen des faits : la moyenne d'âge des sénateurs élus en septembre 2011, inférieure à celle des députés, a suffi à ébranler quelques certitudes bien établies. Quand bien même Quand bien même nous abonderions dans votre sens, que nous laisse suggérer votre logique d'approche à l'égard des sénateurs représentant les Français de l'étranger, si ce n'est si ce n'est qu'ils sont possiblement dépourvus des compétences requises ? Non, rien de tout cela n'est très sérieux et, pour l'heure, rien n'oblige à détenir un mandat pour se porter candidat. Votre argument, monsieur le rapporteur, tombe de lui-même. sur le lien organique entre institution sénatoriale et collectivités territoriales, des choses d'une vérité toute relative ont été dites. Rappelons, à toutes fins utiles, que le Sénat n'est pas « sous un mandat spécifique des collectivités », à l'instar du Bundesrat allemand, tout juste bénéficie-t-il d'une fonction complémentaire reconnue par la Constitution. À la fin des fins cependant, quelle que soit l'issue que le législateur donnera à cette disposition organique, armons-nous d'une seule certitude l'alignement de l'âge d'éligibilité en vertu duquel on est mesure d'élire et d'être élu n'est qu'une faculté qui est donnée ; soyez rassurés, ce sont les grands électeurs qui auront le dernier mot Voilà, pour l'essentiel, les ressorts de notre positionnement qui vous enjoignent à entrevoir dans l'argument des années un facteur discriminant injustifié que le législateur organique gagnerait à abroger. Tâchons aujourd'hui, mes chers collègues, de faire oeuvre utile. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen de la proposition de loi organique déposée par M. Gattolin et certains de ses collègues du groupe LREM a au moins le mérite de nous permettre d'échanger sur la révision constitutionnelle, mise en attente depuis la suspension de son examen par les députés l'été dernier. Faut-il abaisser l'âge d'éligibilité des sénatrices et sénateurs ? le groupe que je préside réitère aujourd'hui une position déjà affirmée en 2003 et 2011, lorsque nous avions proposé nous-mêmes une telle évolution. Je suis assez étonnée de constater la persistance de la majorité sénatoriale dans une attitude crispée de maintien à vingt-quatre ans d'un seuil de maturité pour accéder à l'auguste fonction sénatoriale.

pourquoi persister à afficher que le mandat sénatorial exigerait plus d'expérience que l'exercice de la présidence de la République ? Ce n'est pas sérieux ! Cette crispation n'a aucun fondement constitutionnel. Vous affirmez en effet que le candidat sénateur ou la candidate sénatrice doit avoir exercé un mandat local de six ans pour pouvoir exercer pleinement sa fonction. Ce n'est pas dans la Constitution, et- faut-il le rappeler ? -, si le Sénat assure la représentation des collectivités locales, il ne les représente pas directement. Faut-il rappeler également que nombre de sénatrices et de sénateurs n'ont pas exercé de mandat local et qu'ils n'en demeurent pas moins d'excellents parlementaires ? Car, rappelons-le, le Sénat est une assemblée législative, une assemblée de contrôle de l'exécutif, à l'instar de l'Assemblée nationale. Cette évolution se poursuivra sans doute avec l'adoption du non-cumul des mandats. Être élu ou l'avoir été peut être un atout, la garantie d'une bonne connaissance de certains enjeux, mais être élu ne fait pas tout. Le Parlement manque cruellement, par exemple, de représentants du monde du travail, de représentants des salariés. La lecture du rapport de M. Segouin étonne. À partir de cette question de l'âge et d'un surprenant éloge de la sagesse liée à l'accumulation des années, M. le rapporteur construit une défense inconditionnelle d'un Sénat immuable au rôle perpétuellement positif et garantie absolue de la stabilité de nos institutions.

Vous rappelez les propos du président de la commission des lois, M. Philippe Bas, qui qualifiait le Sénat de « seul pouvoir non aligné, libre et indépendant ». Je sais qu'en politique la coutume est d'avoir la mémoire courte. Mais peut-on affirmer que le Sénat, face à la gauche plurielle de M. Jospin en particulier, et lorsqu'il est en phase avec la couleur politique de la majorité présidentielle, fut et est non aligné ? Oui ! Je ne le crois pas. Le bicamérisme mérite d'être évalué et repensé. Je ne partage pas l'idée d'une nécessaire assemblée modératrice, d'une assemblée freinant les ardeurs du peuple, s'imposant à l'Assemblée nationale du fait de l'élection au suffrage universel direct. Abaisser l'âge d'éligibilité à dix-huit ans ne menace en rien le rôle actuel du Sénat et sa fonction historique. Ce qui est certain, mes chers collègues, c'est que la crise profonde que nous vivons aujourd'hui, une crise profonde de représentation, une crise politique grave, s'appuyant sur un désastre social, avec une croissance forte des inégalités et de l'injustice sociale, exige autre chose qu'un exercice d'autosatisfaction sur les institutions de notre pays. Il faut repenser en profondeur le rapport entre le peuple et les institutions, assurer sa juste représentation. Le Sénat, il est vrai, a parfois joué un rôle positif ces dernières années. C'est la proportionnelle, tant détestée sur les travées de la majorité sénatoriale, qui a pourtant permis au Sénat de préserver, de manière très partielle mais réelle, une forme de débat pluraliste. Ce n'est finalement qu'un sentiment superficiel, car le Sénat accompagne et soutient depuis toujours les projets libéraux, comme récemment la loi ÉLAN ou la réforme ferroviaire. Nous ne sommes oui, pourquoi pas ? Mais dans le cadre d'une vaste réforme constitutionnelle, en rupture avec la logique présidentialiste ! Oui, monsieur Gattolin, nous voterons votre proposition de loi organique, car permettre aux jeunes de siéger au Sénat nous paraît être la moindre des choses. Mais nous ne sommes pas dupes. Votre groupe soutient, bien entendu, le projet constitutionnel de M. Macron. Ce projet, vivement contesté, s'attaque au Parlement et aux droits des parlementaires la diminution du droit d'amendement et une course infinie à l'efficacité, démarche partagée pour l'essentiel, par la majorité sénatoriale, malgré les froncements de sourcils de notre président Larcher. M. Macron propose de réduire fortement le nombre de parlementaires. En quoi abaisser la représentation démocratique sert-il la démocratie ? Nous attendons toujours une réponse à cette question. Croyez-vous, monsieur Gattolin, que le fait de réduire de 30 %, ou même de 20 %, le nombre de parlementaires, permettra à des jeunes d'être élus ? Il y a une part de naïveté, pour rester aimable, à le croire, tant il est évident que la réduction du nombre de sièges favorisera les élus les plus aguerris. Il y a donc une contradiction majeure dans le fait de soutenir les projets profondément antidémocratiques d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et de proposer aujourd'hui d'ouvrir le Sénat à la jeunesse. Nous voterons ce texte par principe, fidèles à notre engagement pluraliste républicain et citoyen. Mais nous le voterons sans illusion, avec clairvoyance et lucidité, car un rude combat s'annonce pour préserver nos institutions de dérives hyper-présidentialistes, voire autoritaires, et pour, au contraire, les ouvrir au peuple, lequel manifeste chaque jour sa colère et son rejet d'un système politique qui le tient à l'écart du pouvoir qu'il est, aux termes de la Constitution-

eu. Ces personnes, qui ont été élues après avoir eu d'autres activités, nous apportent leur expérience, leurs compétences et leur vision des choses. C'est très bien ainsi ! Après tout, dans chaque département, ce sont les électeurs qui votent, et ils votent pour qui ils veulent. Tout le monde peut se présenter,

la moitié du groupe -, je voterai cette proposition de loi, en cohérence avec la position qui était la mienne en 2011 lorsque nous avions débattu de l'amendement de notre ancienne collègue Nicole Borvo Cohen-Seat.

et sa vocation particulière découlant de l'article 24 de la Constitution était de ne pas voter la loi sur le non-cumul.

le choix de l'électeur pourrait être considéré comme réduit lorsqu'un Français jouissant de ses droits civiques est écarté de son droit d'être candidat. C'est une véritable question de fond. D'un autre côté,

l'abaissement de l'âge, qui est intervenu à deux reprises depuis le début de ce siècle, n'a pas vraiment modifié l'âge moyen des parlementaires au Sénat.

faut que nous vivions dans des institutions équilibrées entre l'exécutif et le législatif. L'expérience que j'ai pu acquérir, comme parlementaire ou comme ministre, me fait dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire

La question que soulève sa proposition de loi est très simple : à quel âge peut-on être candidat aux élections sénatoriales ? Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste a mandaté sa plus jeune sénatrice pour

nous sommes à quelques semaines de la reprise des travaux du Parlement sur la révision constitutionnelle. Je rappelle que cette réforme des institutions souhaitée par le Président Macron ne se limite pas à un projet de loi constitutionnelle, mais donnera lieu à l'examen d'un projet de loi organique et d'un projet de loi ordinaire. Autrement dit, nous nous apprêtons à avoir un débat global sur l'architecture de nos institutions, y compris sur le rôle et la composition du Sénat. Avant même de savoir si l'on est pour ou contre ce que nous propose notre collègue, nous devons nous interroger sur l'opportunité d'avoir ce débat aujourd'hui, alors qu'il aurait toute sa place dans le cadre du débat sur la réforme de nos institutions. Selon moi, cette proposition de loi aurait sa place sous forme d'amendement au projet de loi organique que présentera le Gouvernement.

Il me semble important de rappeler, en écho aux propos de notre rapporteur, que le Sénat n'a pas été sourd sur cette question. Il a déjà fait évoluer deux fois cette condition d'éligibilité depuis 2003. C'était nécessaire, et ces évolutions ont été bénéfiques à la Haute Assemblée. Il ne faut donc pas nous faire de mauvais procès, celui d'un Sénat qui serait rigide et hostile par principe à la réforme. Pour Pour autant, cela signifie-t-il qu'il faudrait systématiquement s'aligner sur toutes les évolutions adoptées pour nos collègues députés ? Certainement pas

par l'INSEE. C'est nous qui allons les chercher le jour des élections pour leur dire : « Eh, oh, il faut peut-être aller voter, vous avez été inscrits sur les listes ! » Voilà la réalité !

venir défendre la cause de ma collectivité sans en connaître n'en serait qu'un petit bout

la première ? Le bicamérisme, la différenciation des deux chambres, voilà ce qui est en jeu Pour s'en persuader, il suffit de lire l'article L.O. 296 du code électoral, que l'on nous propose de modifier : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. » Tout est dit ! Si nous supprimons cette condition particulière d'éligibilité, toutes les autres seront les mêmes que pour l'élection des députés. Mes chers collègues, nous sommes tous attachés à la défense de notre assemblée. Pour bien la défendre, nous devons garder en tête un principe simple à la veille du débat constitutionnel : elle ne doit pas devenir un clone de l'Assemblée nationale. Elle doit être différente, sinon, demain, son existence finira par être remise en cause. C'est aussi simple que cela ! Exactement ! Vous l'aurez compris,

Abaisser l'âge d'éligibilité à dix-huit ans rajeunirait-il le Sénat ? Est-il nécessaire de le rajeunir ? Il est vrai que la fonction de sénateur, dans l'imaginaire populaire, ne laisse pas immédiatement entrevoir un jeune de dix-huit mais plutôt un homme, d'un âge certain, d'une certaine corpulence, aux cheveux blancs, ... Et rares ! ... bref quelqu'un de sérieux, soit l'incarnation de l'origine étymologique du mot. Cet Cet imaginaire populaire ne repose pas seulement sur la représentation des dessinateurs de presse ; il s'appuie sur l'histoire de la Haute Assemblée, dont l'ancêtre, sous le Directoire, se nommait le Conseil des Anciens et avait avait vocation, de par sa composition d'une élite âgée- l'âge minimum étant alors de quarante ans -, à contrebalancer les ardeurs des députés, plus jeunes, plus fougueux et plus progressistes. N'est-ce pas encore le cas aujourd'hui ? Pour avoir échangé avec Pierre Cazeneuve, cofondateur du parti politique Allons Enfants et élu municipal de la commune de Saint-Cloud, qui a su convaincre notre collègue André Gattolin de déposer cette proposition de loi, j'entends les arguments qui sous-tendent cette démarche. Le Sénat reste désormais la seule institution à fixer un seuil d'âge minimum au-delà de la majorité. Ainsi, à dix-huit ans, comme cela a été rappelé, on peut être candidat à la présidence de la République, mais pas sénateur. Ainsi les jeunes élus dans nos instances municipales, départementales ou régionales sont forcés, sous peine d'amende, de prendre part à une élection à laquelle ils ne peuvent se présenter. Cette relative absurdité nous permet de prendre conscience que l'implication dans la vie de la cité- la -, tout comme la valeur, n'attend point le nombre des années. Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, près de quarante grands électeurs avaient moins de vingt-quatre ans en septembre 2017. L'objectif recherché- rapprocher les jeunes de la politique et les intéresser au débat public -est louable. Combien serons-nous à déplorer leur faible participation lors des prochaines élections européennes ? Seuls 29 % des dix-huit à vingt-cinq ans s'étaient déplacés en 2009 et 27 % en 2014. Avec une certaine pointe d'humour, Pierre Cazeneuve, dans une interview accordée à le 14 novembre dernier, avançait un argument en faveur du rajeunissement nécessaire de la Haute Assemblée : « Certains sénateurs souffrent de cette image de maison de retraite politique parfois associée au Sénat. » Cet argument est largement illustré, et j'ai avec moi quelques dessins en témoignent. En tant que benjamine de cette institution, je souhaiterais rassurer les plus inquiets : non, d'être dans une maison de retraite ! Non, je n'ai pas fait une entrée accélérée en EHPAD ! Non, je n'ai pas perdu mon énergie et ma vitalité depuis un an ! Très bien ! Je dirai même que l'agenda d'un sénateur n'a rien à envier à celui d'un ! je me sens parfaitement bien intégrée dans cette institution. Certes, je suis peut-être parfois un peu en décalage avec mon prisme de raisonnement qui peut emprunter aux caractéristiques de la génération X ou mes contraintes de jeune mère de famille. Pour autant, j'ai le sentiment de poursuivre les mêmes objectifs que l'ensemble de mes collègues : défendre et promouvoir mon territoire, mes valeurs et mes idées, tout en gardant à l'esprit l'intérêt général et l'équilibre républicain. Aurais-je pu le faire à dix-huit ans, tout juste sortie du lycée ? Je ne le crois pas. Devenir un législateur ne s'improvise pas. Cela s'apprend au gré de ses études et de ses expériences professionnelles et électives.

Pour représenter, il faut connaître, avoir expérimenté, mis les mains dans le cambouis. L'âge de vingt-quatre ans permet d'avoir à son actif un mandat complet d'élu local au moment de la candidature. De même qu'« on ne naît pas femme, on le devient », ... Simone de Beauvoir ! ... on ne naît pas sénateur, on le devient. Avant de conclure, je remercie André Gattolin et Pierre Cazeneuve d'avoir illustré avec cette proposition de loi l'implication d'une partie de notre jeunesse dans le fonctionnement de nos institutions. Il appartient aux partis politiques institutionnalisés de se donner les moyens d'écouter cette jeunesse qui ne manifeste pas, ne se révolte pas, mais veut proposer et agir pour son avenir et celui de ses enfants. Je pense cependant qu'il ne faut pas aller trop vite

et à fixer l'entrée en vigueur de cette modification au prochain renouvellement sénatorial. Historiquement, l'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales est plus élevé qu'aux élections législatives.

Trois éléments au moins viennent apporter un éclairage sur cette particularité sénatoriale. Tout d'abord, l'existence d'un âge d'éligibilité plus élevé pour les sénateurs résulte d'un compromis initial, après la Révolution française, puis sous la III République, pour concilier évolution du régime et pacification sociale. Ensuite, l'âge est perçu comme un facteur de modération. Enfin, l'âge d'éligibilité plus élevé pour les sénateurs reflète la valorisation de l'expérience au sein des collectivités territoriales. En effet, ce seuil d'éligibilité a été défini pour permettre aux sénateurs d'acquérir une expérience locale avant d'entrer au Palais du Luxembourg. Ce débat relatif à l'alignement de l'âge d'éligibilité des sénateurs sur l'âge de la citoyenneté, s'il n'est pas nouveau, ne peut pas avoir lieu en dehors du cadre de projets plus larges. Il apparaît en effet bien plus opportun et pertinent que ce sujet soit examiné dans le cadre des débats à venir sur les réformes institutionnelles et l'avenir du bicamérisme. En outre, à l'échelle internationale, l'âge d'éligibilité est généralement plus élevé dans les chambres hautes que dans les chambres basses. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à ce jour, rien ne justifie raisonnablement la nécessité de procéder une nouvelle fois à l'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs.

C'est donc une expérience minimum requise dont le caractère paraît évident, et je ne vois rien ici qui ressemble, de près ou de loin, à une « justification assez floue », comme l'avancent imprudemment nos collègues Marcheurs. C'est même, bien au contraire, pleinement cohérent avec la mission de représentation des collectivités territoriales confiée au Sénat, depuis soixante ans, par la Constitution. Fondamentalement, les deux assemblées françaises ne sont pas identiques, mais elles se complètent parfaitement. Notre mode de fonctionnement assure même la continuité de l'État, et ce n'est pas là un détail. Si nos institutions donnent clairement la primeur dans les décisions finales à l'Assemblée nationale et à nos collègues députés qui y siègent, le Sénat jouit, lui, d'une spécificité incontournable et révélatrice de sa sagesse légendaire. En effet, le Sénat, à la différence de l'Assemblée nationale, est une assemblée permanente. Le chef de l'État ne peut donc pas la dissoudre. C'est précisément pour ces raisons, notamment, que la réforme constitutionnelle ourdie par le Président de la République est dangereuse, puisqu'elle conduit, ni plus ni moins, à une dissolution déguisée du Sénat. Vouloir aligner la limite d'âge requis pour devenir sénateur sur celle exigée pour devenir député, c'est ignorer totalement l'essence même du bicamérisme. Oui, la jeunesse incarne l'avenir Mais est-ce à dire que les aînés ne doivent pas être écoutés ? Est-ce à dire que la fougue de la jeunesse doit être élevée au rang d'alpha et d'oméga démocratique ? Je n'en crois rien Je suis convaincu, bien au contraire, que l'expérience est un trésor dont nul ne peut se passer. Il n'est qu'à parcourir le Palais du Luxembourg et son histoire pour s'en persuader.

la tempérance vient avec l'âge. Je ne goûte pas forcément les comparaisons internationales, mais c'est précisément pour cette raison de tempérance qu'un pays jeune comme les États-Unis place l'âge minimal à trente ans pour devenir sénateur. Et que dire alors de nos voisins et amis Italiens

cette limite d'âge ne crée aucune injustice, contrairement à ce que vous avancez. Elle n'empêche en rien un Français de dix-huit ans désirant s'engager pour la Nation en exerçant un mandat parlementaire, d'être candidat à un siège de député. Si nos collègues Marcheurs veulent faire oeuvre utile, qu'ils commencent par faire en sorte que l'ensemble des jeunes Français de dix-huit ans sachent réellement ce que sont nos institutions. Une interrogation écrite donnerait, j'en ai bien peur, des résultats très contrastés. Ça, c'est une anomalie ! Je serais donc surtout partisan de baisser l'âge requis pour connaître réellement les institutions de notre pays. Si nous accueillons régulièrement autant de jeunes collégiens ou lycéens au Sénat, c'est bien pour cette raison. Décidément, avec cette proposition de loi organique de nos collègues du groupe La République En Marche, le nouveau monde défend, une fois encore,

et, lorsque le bicamérisme s'imposa, la question de la composition différenciée de la chambre haute se posa. Tantôt chambre honorifique pour une noblesse déchue de ses privilèges sous la Restauration, tantôt haut lieu des soutiens issus de tous horizons du régime bonapartiste, l'enjeu fut toujours de savoir comment choisir cette seconde chambre et quelle légitimité lui donner. Mode d'élection, âge et conditions d'éligibilité, notre pays a donc cherché dès les origines du système parlementaire puis de la République parlementaire à différencier les deux chambres. C'est bien cette différenciation qui est la raison d'être du Sénat. Tout d'abord, dans un pays fortement centralisé, le Sénat républicain s'est imposé, par son mode d'élection, comme la chambre des territoires, et il a toujours contrebalancé la vieille passion française pour le jacobinisme. En cela, il porte une vision qui enrichit encore les débats et l'action publique tout en étant pleinement l'une des deux chambres du Parlement. Le Sénat est aussi par son propre calendrier une voix dissemblable. C'est essentiel depuis la réforme du quinquennat et l'élection quasi simultanée du Président de la République et des députés. Enfin, grâce

Ce rapport est parfois source de sarcasmes, alors que nous vivons aujourd'hui sous l'injonction permanente du mouvement ; ce temps long est pourtant la clef pour dépassionner. Le législateur spartiate Lycurgue le disait déjà : « Il rassembla ce conseil de sénateurs [ ...] et donna pied ferme et assuré à l'État. Donner pied ferme et assuré à l'État, telle est l'identité du Sénat. Cette identité particulière a notamment pour origine le mode d'élection et l'âge minimal d'éligibilité des sénateurs. Certes, en 2011, ce qui caractérisait le Sénat par rapport à l'Assemblée nationale du point de vue des conditions d'éligibilité et d'élection a déjà été atténué, et je ne suis pas sûr que ce fût une bonne chose. La solution d'un écart d'âge théorique d'un citoyen ayant effectué au moins un mandat local est à mon sens la plus raisonnée. Bien évidemment, elle n'est pas, de mon point de vue, parfaite, puisque je suis de ceux qui auraient préféré que le législateur fixe une barre plus haute. Toutefois, dans une chambre des territoires, comment penser, au minimum, défendre les collectivités locales sans les connaître et sans avoir déjà exercé au moins un mandat ? Comment se prévaloir des qualités de recul et d'analyse sans instaurer ce seuil d'âge minimal ? Ce seuil n'a pas empêché l'âge moyen du Sénat d'être assez proche de celui de l'Assemblée nationale. Il n'a pas non plus empêché un sénateur de l'Essonne, qui n'était pas encore le chef de file des Insoumis, d'être l'un des plus jeunes sinon le plus sage des sénateurs de France. J'en viens à l'âge d'éligibilité du Président de la République, argument massue de nos collègues Sueur et Gattolin. Pour justifier votre proposition de loi organique, monsieur le sénateur Gattolin, vous proposez d'abaisser l'âge d'éligibilité des sénateurs pour l'aligner sur celui du Président de la République, dont, vous en conviendrez, la sagesse et le recul doivent être exemplaires, plus encore que, certainement, que ceux des sénateurs, eu égard aux responsabilités qu'il assume. Alors, pourquoi plutôt aligner l'âge minimal d'élection du Président de la République sur celui des sénateurs, afin de contribuer théoriquement à ce qu'il fasse montre des mêmes qualités Je sais combien tout ce que je viens de dire est difficile à entendre dans une société de l'immédiateté ; je sais qu'il est difficile, dans notre société, de comprendre que l'expérience peut donner des droits supplémentaires ; je sais qu'il est passé de mode de justifier le bicamérisme différencié en puisant des arguments dans l'histoire ; mais, franchement, au-delà des difficultés de notre époque à accepter les leçons du passé, cette tendance qui vise peu à peu à réduire ce qui différencie les deux chambres n'entre-t-elle pas dans la logique qui cherche à gommer aujourd'hui la différenciation entre les chambres, puis, le jour où les deux chambres se ressembleront, à dire qu'il y en a une de trop ? Je suis persuadé que, ce jour-là, la démocratie aura reculé ; pour l'instant je m'en tiendrai à

Aujourd'hui, le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un mandat local non exécutif. L'amendement n° 7 rectifié de M. Mézard tend à supprimer cette incompatibilité pour les suppléants de sénateur ou de député, d'entre eux sont contraints de quitter leur mandat local pour siéger au Parlement, parfois de manière brève. On comprend la logique de cet amendement, mais celui-ci dépasse largement le champ de la présente proposition de loi organique.

jeune et avoir des problèmes d'audition ... Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.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

Or, pour les citoyens, il est justement incompréhensible que des personnes dont le casier judiciaire mentionne des condamnations pour corruption puissent devenir sénateurs. Cette remarque vaut aussi pour des délits du même type, comme la prise illégale d'intérêts ou le blanchiment et,, pour des crimes ou des délits d'atteinte à la personne : homicides, violences graves

Je précise que celui-ci n'a pas un objectif répressif contre les individus, mais qu'il vise la protection de l'exercice du mandat de parlementaire, à l'instar de ce qui existe dans de nombreuses professions ou fonctions. Je précise également que la mention d'une condamnation figurant au casier judiciaire n'est pas toujours définitive. Indépendamment de la réhabilitation, l'inscription au casier judiciaire peut être écartée par le juge, soit au moment du jugement, soit, si la demande lui en est faite. L'amendement n° 1 rectifié de M. Cabanel tend à imposer un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections législatives et sénatoriales. Cela remplacerait donc les peines d'inéligibilité qui sont prononcées au cas par cas par le juge. Ce débat existe depuis plusieurs années. Nous partageons un objectif commun : garantir la probité de la vie politique. Toutefois, le Parlement a rejeté cet amendement à de nombreuses reprises, car celui-ci soulève des difficultés sur le plan constitutionnel. En juillet 2017, la garde des sceaux a clairement rappelé que ce dispositif pouvait être assimilé à une peine automatique. Certes, il est applicable aux concours de la fonction publique, mais le droit fondamental d'exercer un mandat électif va au-delà de la carrière professionnelle. pour la confiance dans la vie politique a déjà prévu un mécanisme, déclaré conforme à la Constitution : l'instauration d'une peine d'inéligibilité obligatoire pour certains crimes et délits, sauf décision contraire du juge. Le Sénat avait d'ailleurs complété ce texte en y ajoutant le harcèlement sexuel ou moral, l'escroquerie en bande organisée, l'association de malfaiteurs et l'abus de biens sociaux. Enfin, le dispositif proposé au travers de cet amendement serait moins efficace que le droit en vigueur. En effet, une mention sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être effacée six mois après la condamnation certains condamnés pourraient ainsi obtenir la radiation de cette mention et d'autres non, sans que l'on puisse s'assurer de la cohérence de ces décisions. Nous aurons certainement ce débat à l'occasion des réformes institutionnelles.

L'amendement n° 4 rectifié de M. Joyandet tend à supprimer l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la présidence du conseil de surveillance d'une entreprise nationale ou d'un établissement public national. amendement n° 5 rectifié est un amendement de repli : il concerne uniquement la présidence du conseil de surveillance d'un établissement public de santé. Dans une décision du 12 avril 2018, le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu'un sénateur ne pouvait pas être vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris- les parlementaires peuvent toutefois rester membres du conseil de surveillance sans en assurer la présidence. Cette jurisprudence est particulièrement complexe, je le conçois, et il y a sans doute des marges de progression. Un toilettage serait certainement opportun concernant ces incompatibilités à titre d'exemple, nous pourrions nous interroger sur l'interdiction pour un parlementaire membre du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement. Ces questions pourraient être abordées lors des prochaines réformes institutionnelles, mais, en l'état, elles dépassent le champ de la proposition de loi organique, que la commission propose d'ailleurs de ne pas adopter. La commission demande donc le

nous ne sommes plus maires, nous ne sommes plus présidents de conseil départemental, nous ne sommes plus rien. Nous ne pouvons même pas présider bénévolement le conseil de surveillance d'un hôpital local, quand bien même ce dossier

Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l'article 2, je vous rappelle que, si celui-ci n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi organique, dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explications de vote sur l'ensemble.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande